chers collègues, au nom du Bureau du Sénat, j'appelle chacune et chacun d'entre vous à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat le respect des uns et des autres, ainsi que celui du temps de parole pour permettre à chaque collègue de bénéficier de la diffusion complète de sa question et de la réponse. La parole est à M. David Assouline, pour le groupe socialiste et républicain. Madame la ministre, dans ce monde où les médias ont un impact profond et quotidien sur la vie de nos concitoyens, et dans un contexte où la révolution technologique bouleverse tous les formats,

Nous devrions vite organiser non pas un Grenelle, mais un Valois de l'audiovisuel, avec pour priorité le service public : notre devoir est de lui donner les moyens d'être fort et créatif et de répondre à ses missions d'intérêt général grâce à des programmes de qualité. Cette année, l'État manque à sa parole en privant France Télévisions de 79 millions d'euros. Mais ce qui nous inquiète encore davantage, c'est le document budgétaire qui a « fuité » de votre ministère et qui, sous couvert de synergie,

je vous remercie pour cette question qui me donne l'occasion de m'exprimer clairement et solennellement devant la représentation nationale sur le sujet de l'audiovisuel public. Comme je l'ai déjà dit, le document que vous évoquez et qui a été rendu public n'est pas une ébauche de stratégie, mais un exercice de recensement des pistes mises sur la table ces dernières années ... Rien à voir ! ... par divers rapports, notamment des rapports parlementaires issus de votre Haute Assemblée ou de la Cour des comptes. Il s'agit donc d'un document provisoire

j'ai demandé des contributions aux sociétés de l'audiovisuel public en parallèle du travail réalisé par les administrations. Ces contributions nous sont parvenues et montrent une vraie volonté d'avancer. Je les en remercie ! Dès demain, je recevrai d'ailleurs individuellement chaque dirigeant pour échanger sur ces propositions.

Demain, si l'audiovisuel public veut continuer à jouer un rôle central de média universel et populaire, il doit offrir une vraie alternative. Je veux rappeler et saluer ici la force et les singularités des médias de service public, lesquels assurent une information de référence dans un univers où circulent les fausses nouvelles, un investissement déterminant dans la création et dans les formats originaux, proposent une offre globale qui doit s'adapter au numérique, et traduisent une volonté de s'adresser à la jeunesse et de contribuer au rayonnement international de la France

et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes. Madame la ministre, le ministre de l'agriculture a participé au conseil interministériel de la mer réuni vendredi dernier à Brest par le Premier ministre. pour saluer l'intérêt du Gouvernement pour les problématiques liées à la mer et aux océans, qui représentent une opportunité majeure pour l'économie et le développement durable de notre pays. Néanmoins, comme vous le savez, le 27 novembre prochain, les marins pêcheurs français ont décidé de bloquer le port de Calais pour protester contre l'usage de la pêche électrique près de nos côtes, notamment de la part de navires hollandais. Ces derniers profitent d'une dérogation incompréhensible au droit de l'Union européenne, qui interdit en principe la pêche électrique. L'action des pêcheurs français est un signal fort de leur détresse face à une pratique qui détruit de manière massive et sans distinction les stocks de poissons, met en péril leur reproduction et a des conséquences désastreuses sur l'environnement. Il y a quelques jours, mon collègue député Paul Christophe a attiré l'attention du ministre de l'agriculture sur cet enjeu majeur pour l'avenir de la filière des produits de la pêche maritime. de la pêche électrique révèle les dilemmes de la politique commune de la pêche au niveau européen. Elle apparaît tiraillée entre, d'un côté, une gestion durable des ressources halieutiques et, de l'autre, un déficit commercial abyssal en matière de produits de la mer. Madame la ministre, avec précision la position que la France entend défendre au niveau européen pour concilier protection de l'environnement, autosuffisance et revenus décents pour les pêcheurs français. Je souhaite ajouter que le niveau européen sera crucial pour traiter la question du Brexit. Ce sont les pêcheurs français, de Bretagne et des Hauts-de-France notamment, qui auraient le plus à perdre si le Royaume-Uni fermait l'accès à ses eaux territoriales. Nous espérons que vous porterez les inquiétudes de la filière au niveau européen dans vos échanges

la pêche au chalut électrique est interdite dans l'Union européenne. Cependant, comme vous l'avez relevé, les règles communautaires prévoient des dérogations pour un nombre limité de navires : au maximum 5 % des chaluts à perche par État membre. En mars 2016, la Commission européenne a proposé de supprimer cette limitation ; la France s'y est fermement opposée au conseil des ministres de l'agriculture et de la pêche du 11 mai 2017. En l'état actuel de nos connaissances et faute d'évaluation précise de son impact sur les stocks de poissons et sur l'environnement, ce mode de pêche doit rester strictement limité. Le Gouvernement continuera donc à défendre cette position dans les discussions engagées avec le Parlement européen. Le ministre de l'agriculture Stéphane Travert évoquera, quant à lui, cette question avec son homologue néerlandaise lors du conseil des ministres de l'agriculture des 11 et 12 décembre prochains. Permettez-moi enfin de rappeler que le Gouvernement est mobilisé pour défendre les intérêts des pêcheurs français, qu'il s'agisse des négociations du Brexit ou de la future politique commune de la pêche après 2020. Comme l'a dit le Premier ministre, le secteur de la pêche fait partie de nos priorités dans la négociation sur le retrait du Royaume-Uni Nous soutenons Michel Barnier qui mène cette négociation. Les échanges débuteront dès que le Conseil européen estimera que des progrès suffisants ont été accomplis sur la première phase des discussions avec les Britanniques. Nous sommes par ailleurs déterminés à travailler dans le sens d'une amélioration de la politique commune de la pêche, qui peut et qui doit concilier protection de l'environnement et niveau de vie décent pour nos pêcheurs, comme vous le demandez

qui ne relève en rien d'une stratégie globale et qui n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les élus locaux ! Sa conséquence directe est la mise à mal d'un grand nombre de bailleurs sociaux, mais aussi de collectivités locales, dans la mesure où ces dernières sont engagées par les garanties d'emprunts. La ponction que vous souhaitez effectuer sur les organismes aura un impact sur les constructions nouvelles, l'entretien du parc existant et la rénovation. Les élus locaux ont le sentiment que cette mesure n'a d'autre raison d'être que de trouver une

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, je vous remercie de cette question, à laquelle je réponds bien volontiers. Je salue votre engagement sur ce sujet, ainsi que celui de la sénatrice et du sénateur que vous avez bien voulu associer à votre question.

La cathédrale, c'est la réforme du logement que le Gouvernement proposera, que le Parlement discutera et qu'il nous faut préparer. La porte d'entrée, c'est la volonté clairement exprimée et parfaitement assumée de faire en sorte que le montant des crédits budgétaires affectés aux aides personnalisées au logement diminue

J'ai fait un certain nombre de propositions aux organismes de logement social, notamment celle d'associer à la baisse des crédits budgétaires une éventuelle augmentation de la TVA qui pèse sur le logement social, afin d'éviter d'affecter trop durement leurs recettes d'exploitation. J'ai proposé des contreparties importantes : plus de 6 milliards d'euros pour le logement social ! Cette somme permettrait d'accompagner les efforts d'investissements à l'avenir. Autrement dit, notre plan est très complet, et je crois que vous le savez, madame la sénatrice. Je crois que tous ceux qui regardent ce sujet avec attention le savent. Les discussions sont en cours

que vont frapper nos concitoyens mal logés du quartier de Caucriauville, pas à la porte de Matignon ! La parole est à Mme Sophie Joissains, pour le groupe Union Centriste. Madame la présidente, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur. Ces dernières semaines ont été tragiques pour les policiers et les gendarmes. Une vague de suicides a touché nos forces de sécurité, ce qui ne peut bien entendu pas nous laisser indifférents. Après un pic en 2014, année noire au cours de laquelle cinquante-cinq policiers et une trentaine de gendarmes avaient mis fin à leurs jours, le taux de suicide parmi les forces de l'ordre a décru en 2015 et 2016. Cela ne sera malheureusement pas le cas cette année. Le métier qu'exercent policiers et gendarmes au quotidien n'est pas un métier comme les autres, car ceux-ci sont évidemment régulièrement confrontés à la mort, à la violence, ainsi qu'à la misère humaine. Le stress que subissent nos forces de sécurité- gendarmes et policiers confondus -depuis la mise en place de l'état d'urgence a accru le malaise et parfois la détresse dans leurs rangs. L'ampleur du risque terroriste, la violence quotidienne et, enfin, le manque de reconnaissance, voilà ce qui use policiers et gendarmes ! Il y a aussi, comme le pointe un syndicat, le manque d'effectifs : « 70 % des forces de police expliquent ne plus pouvoir faire face à leur charge de travail ». Le même syndicat dénonce aussi l'existence de formations parfois considérées comme inadaptées ou trop courtes. votre prédécesseur avait annoncé un plan de prévention qui prévoyait notamment le recrutement de psychologues ou la refonte des cycles de travail. Quasiment trois ans après, la situation se dégrade à nouveau dans de larges proportions : qu'en pensez-vous ? Ces mesures ont-elles été effectivement mises en oeuvre ou se sont-elles révélées inefficaces ? La parole

il est toujours difficile d'expliquer de tels gestes dont les raisons sont multiples, dont les causes sont complexes. Si ce sont souvent des raisons intimes,

Ils doivent en effet maintenir l'ordre public, sont amenés à lutter contre le terrorisme, traquent les criminels et les délinquants, et sont donc confrontés à la violence, ainsi qu'à la part la plus sombre de notre société. Oui, cela peut mener à une tension et à un stress extrêmes. C'est pourquoi, pour répondre précisément à votre question, nous avons renforcé le soutien psychologique par l'embauche de psychologues cliniciens, aussi bien dans la police nationale que dans la gendarmerie nationale. Nous avons également développé une politique de sensibilisation personnalisée des élèves dans les écoles de gendarmerie et de police.

! La parole est à M. Michel Amiel, pour le groupe La République En Marche. Madame la présidente, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie et des finances et concerne les difficultés de la filière sidérurgique et l'actualité de la société Asco Industries. Alors que la filière de l'aciérie a connu de nombreuses difficultés ces dernières années, le cas de la société Asco Industries est particulièrement criant. Plombé par une dette de 360 millions d'euros, le groupe Ascométal a été placé en redressement judiciaire le 7 mars 2014. Le tribunal de commerce de Nanterre a choisi un mois plus tard l'offre de reprise du groupe français, portée à l'époque par Frank Supplisson, ancien directeur de cabinet d'Éric Besson, ministre de l'industrie, et par l'industriel Guy Dollé, ex-directeur général d'Arcelor. Aujourd'hui, ce projet bat de nouveau de l'aile et Asco Industries, cette société qui compte 1 500 employés et qui a contracté une dette de plus de 40 millions d'euros, cherche à nouveau un repreneur. La société vient d'être déclarée en cessation de paiement et placée en redressement judiciaire, ce qui lui permettra évidemment de négocier au mieux avec d'éventuels repreneurs. D'ailleurs, un article du journal faisait état d'au moins trois sociétés européennes qui auraient déposé une lettre d'intention. Alors que la situation semble s'enliser une fois de plus, les salariés d'Ascométal risquent tout simplement de perdre leur emploi. De plus, de nombreuses entreprises fournissant des matières premières vont se retrouver en grande difficulté, risquant même jusqu'au dépôt de bilan.

je souhaiterais donc connaître votre position et vos engagements face à une situation qui, à force de se répéter, met un pan entier de notre économie en danger ! La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Amiel, je connais bien les difficultés que rencontre le groupe Ascométal. Soyez assuré que les services du ministère de l'économie et des finances, ainsi que mon cabinet, y sont évidemment très attentifs.

Depuis la reprise à la barre du tribunal en 2014, Ascométal n'a malheureusement pas retrouvé le chemin de la rentabilité. Ce producteur d'aciers longs spéciaux à destination de l'automobile et de l'industrie, notamment du pétrole et du gaz, continue d'enregistrer des pertes massives. Dans ce contexte, face aux besoins de financement pour opérer le redressement du groupe, il a été décidé il y a plusieurs mois d'engager une recherche de repreneurs pour l'ensemble du groupe.

Hier, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit du groupe, qui répond à l'impasse de trésorerie à laquelle il faisait face à court terme. Cette décision devrait donner du temps et permettre de retrouver un cadre favorable à la reprise, ce qui est assez décisif en cours vise donc à organiser une cession ordonnée d'Ascométal, facilitée par l'existence d'un travail en amont sur cette possible reprise. Nous avons un calendrier clair pour déposer une offre de reprise, qui sera par ailleurs fixé dans les jours qui viennent. Pour que la reprise soit

je vous remercie de rappeler que vous n'oublierez pas non plus les sous-traitants ni les fournisseurs. La parole est à Mme Josiane Costes, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Madame la présidente, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice. Les mineurs en danger sont pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance ou, dans les cas de délinquance avérée, par la Protection judiciaire de la jeunesse. Les missions des uns et des autres visent à favoriser l'intégration sociale, scolaire et professionnelle des jeunes et, dans les cas les plus graves, à protéger la société contre des exactions qu'ils pourraient commettre. Qu'ils soient placés en famille d'accueil ou dans un établissement, l'investissement des équipes éducatives est remarquable et les résultats sont globalement positifs. Toutefois, à 18 ans, ils doivent brutalement quitter les structures et retrouver leur milieu d'origine. Les risques de replonger dans la délinquance, voire parfois dans la radicalisation, sont avérés. Il s'agit là d'un gâchis tant sur le plan humain que sur le plan financier, lorsque l'on sait, par exemple, qu'une journée en centre éducatif fermé coûte environ 570 euros par jeune Ne pourrait-on pas envisager un accompagnement transitoire, afin que la sortie des dispositifs soit moins brutale ? Cette sortie ne pourrait-elle pas se faire de façon plus progressive, de manière à davantage consolider les améliorations constatées dans le ? La parole est à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, je vous remercie de votre question. Je vous sais très attentive à un sujet que vous traitez- me semble-t-il -dans le cadre de votre rapport budgétaire. Effectivement, il existe actuellement plusieurs dispositifs pour accompagner les jeunes dans ces temps un peu délicats de rupture, que ce soit le passage à la majorité ou la sortie

pour une durée qui dépasse la majorité. Elle permet ainsi, avec l'accord du jeune, de poursuivre le placement et de continuer la mesure d'accompagnement éducatif. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle favorise le développement de ces mesures en autorisant les tribunaux pour enfants à prononcer cumulativement une peine et une mesure éducative. Dès lors, un jeune qui a commis des faits suffisamment graves pour justifier une sanction pénale pourra également bénéficier de la continuité de son placement dans des établissements relevant de la Protection judiciaire de la jeunesse, qu'il s'agisse d'une structure de type foyer ou d'une autre structure.

Malgré ces dispositifs, les ruptures sont encore trop nombreuses. C'est pourquoi la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant propose aux conseils départementaux de signer des conventions avec les services de l'État pour accompagner ces jeunes. J'ai moi-même demandé à la

groupe communiste républicain citoyen et écologiste. La France, avec d'autres pays européens, s'était donné l'objectif de construire « l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde » en augmentant ses dépenses en matière de recherche et d'enseignement supérieur. Le but était de rattraper notre retard structurel en profitant de l'effet de levier avéré des investissements dans ces domaines. Près de vingt ans plus tard, ce grand dessein a été abandonné, et notre pays demeure toujours dans le bas des classements des dépenses par étudiant et de proportion de titulaires de doctorats. La démographie relativement dynamique de notre pays va accroître le nombre de bacheliers d'environ 35 000 pendant une dizaine d'années. Cet apport précieux aurait pu être mis à profit par le Gouvernement pour tenter de redresser notre situation dans le domaine de la connaissance. Malheureusement, obnubilés par le dogme de la réduction de la dépense publique, vous ne concevez cette masse supplémentaire d'étudiants que comme un trop-plein fâcheux qu'il faut administrer sans frais supplémentaires. Vous avez donc décidé de détourner une partie de ce flot des universités en donnant à celles-ci la possibilité de le filtrer. Dans notre pays, seule la moitié des formations est librement accessible. Vous venez de prendre la grave décision de diminuer encore cette proportion, au risque de jeter sur le marché de l'emploi de nombreux jeunes sans formation. Ce terrible choix, vous ne l'assumez pas directement, vous le reportez sur les universités dans des conditions d'impréparation qui inquiètent élèves, parents et professeurs les risques sont grands d'aboutir à une rentrée universitaire encore plus chaotique que la précédente ... Alors qu'il en est encore temps, nous vous le disons solennellement : renoncez à votre projet, ayez confiance en notre jeunesse et donnez-lui les chances de sa réussite !

terminales2017-2018.fr, qui existe, donne les bons conseils. Dès maintenant, nous programmons, au travers du projet de loi de finances pour 2018, la création de nouveaux BTS, qui permettront à des bacheliers professionnels de réussir leur insertion professionnelle au lieu d'être en échec. Il y a ainsi, à la fois,

La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour le groupe socialiste et républicain.

Nous avions été choqués par les images de ce petit garçon, Aylan, retrouvé sans vie, face contre terre, sur une plage turque. Nous voilà à nouveau confrontés à l'inadmissible : les enquêteurs de l'ONU et plusieurs médias ont mis en lumière des cas d'esclavage en Libye. Concrètement, il s'agit d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont vendus aux enchères comme du bétail sur les marchés libyens. Ne faisons pas semblant de le découvrir, nous le savions tous. Depuis des années, les ONG nous alertent ; leurs derniers rapports de 2016 faisaient état de 45 millions de femmes, d'hommes et d'enfants asservis ; 45 millions, chers collègues ! C'est l'équivalent de la population espagnole cent soixante-dix ans, la France abolissait l'esclavage. Voilà seize ans, sur ces travées, nous adoptions la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Pourtant, ces camps, financés par l'Europe, se développent désormais, avec notre aval, dans des conditions qui constituent un véritable scandale humanitaire. Familles séparées, viols, torture, surpopulation, conditions sanitaires déplorables, tel est le quotidien de ces réfugiés, et, lorsqu'ils parviennent à échapper à ces camps, ils se noient dans la Méditerranée.

Le temps de l'indignation doit maintenant laisser la place au temps de l'action. C'est pourquoi la France, pays des droits de l'homme, doit porter un message fort, qui fera honneur aux valeurs qui nous unissent. Monsieur le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères a indiqué que la France avait demandé une réunion expresse du Conseil de sécurité de l'ONU. et l'Afrique aura également lieu dans cinq jours à Abidjan. Pouvez-vous, dès lors, nous préciser quelle sera la position de la France visant à mettre fin à ce marchandage de vies humaines ?

vous avez raison, ce que nous avons vu, les images diffusées montrant la traite d'êtres humains en Libye, est inadmissible. Vous avez raison, il s'agit d'un crime contre l'humanité ; d'ailleurs, le Président de la République a qualifié cette Vous avez aussi raison de rappeler que, hier, Jean-Yves Le Drian a appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies. La France, terre de droits de l'homme, prend ses responsabilités de membre permanent du Conseil de sécurité, pour porter ce drame humain au plus haut niveau. En revanche, je ne vous rejoins pas lorsque vous parlez de camps financés par l'Union européenne, car ce n'est pas le cas. L'Union européenne vient en aide au HCR et à l'Organisation internationale pour les migrations, pour faire en sorte d'améliorer la vie et le traitement des migrants dans ce pays, la Libye, qui ne connaît pas d'État stable et encore moins de respect des droits de l'homme. Ce que nous faisons en outre, à titre bilatéral, est que nous nous rendons au Niger et au Tchad pour examiner, sur le continent africain lui-même, la situation de ceux qui ont un besoin évident de protection, afin que ceux qui bénéficieraient manifestement du droit d'asile puissent rejoindre directement l'Europe. Ce que nous faisons également nous multiplions les efforts pour que la situation en Libye se stabilise. Nous ne pourrons traiter un problème de cette ampleur- l'Organisation internationale pour les migrations a parlé de 300 000 migrants en Libye et certaines estimations

Depuis 2014, le Sénat s'est engagé dans une ambitieuse action de simplification des normes, en particulier de celles qui sont applicables aux collectivités. Je n'en décrirai pas toute l'ampleur, mais je rappellerai simplement notre dernière initiative : une proposition

en ce sens a d'ailleurs été réitérée hier dans cet hémicycle, mais nous restons toujours sans réponse. Je profite donc de cette période rare où le Gouvernement s'intéresse aux collectivités locales pour vous demander, dans un premier temps, ce que vous envisagez de faire pour répondre à la frénésie normative

permettez-moi de saluer la proposition de loi que vous avez évoquée, qui a été effectivement adoptée à l'unanimité par votre chambre, il y a peu.

Ces villes et ces villages ne sont plus identifiés comme devant bénéficier de cette incitation à l'investissement privé locatif aidé, aux logements intermédiaires ou au prêt à taux zéro, le PTZ.

211 communes classées en zone B2 sortiront du dispositif. La ville de Calais en fait partie, et ce n'est pas une bonne nouvelle dans le contexte migratoire qui l'agite et qui fait fuir les investisseurs de tous ordres.

que restera-t-il à ces communes pour maintenir leur dynamisme, d'autant que leur budget diminué limite leurs marges de manoeuvre ? J'ai le sentiment, monsieur le ministre, que priver ces territoires de cette potentialité ne fera que les isoler davantage dans leurs difficultés et que cela accentuera leurs déséquilibres, ainsi

à taux zéro et le dispositif Pinel. Vous le savez, on a décidé de prolonger ces dispositifs, notamment le prêt à taux zéro, y compris dans les zones détendues- ces fameuses zones B2 et C, que vous avez évoquées dans votre question.

qui prendra du temps, mais c'est le sens de l'histoire et c'est ce vers quoi il faut avancer.

Monsieur le secrétaire d'État, la France et le Cambodge entretiennent des relations extrêmement étroites et privilégiées ; c'est le fruit d'une histoire commune. En particulier, durant le terrible régime des Khmers rouges et le génocide, la France a accueilli des

France, les accords de Paris, qui ont permis à la fois le retour à la paix, le développement économique du pays et un processus de transition vers l'État de droit. de la semaine passée, le régime usé du Premier ministre Hun Sen, au pouvoir depuis trente-deux ans, a procédé à un véritable putsch institutionnel, une cour suprême à sa botte, en supprimant purement et simplement le Parti du sauvetage national du Cambodge, principale force d'opposition.

Pour autant, les États-Unis, le service européen pour l'action extérieure et, très récemment, la Suède viennent de décider d'engager des sanctions. Aussi, face à cette situation,

de Paris et garante des accords en cas de violation de ceux-ci, entend convoquer prochainement la vingtaine d'États qui en sont parties prenantes, afin de persuader le Cambodge et son gouvernement de revenir sur la voie de la démocratie ? La parole

L'arrestation de M. Kem Sokha et l'absence probable de ce parti pour les prochaines échéances sont très préoccupantes. Dans ce cadre, la France est naturellement soucieuse d'être particulièrement mobilisée et présente. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères s'en est entretenu très directement avec son homologue, M. Prak Sokhonn, le 20 novembre dernier, à l'occasion du sommet de l'ASEM. Dans les prochains jours, je réitérerai de notre préoccupation, à l'occasion de la conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie, dont le Cambodge est membre, puisque nous partageons, dans cette instance, un certain nombre de valeurs communes et que nous devons les appliquer. Enfin, dans le cadre européen, il va de soi que le régime préférentiel accordé

votre question, la contribution des sénateurs à la diplomatie parlementaire et au respect des libertés publiques. C'est une caractéristique constante de la Haute Assemblée, et nous savons donc que nous avons votre soutien entier.

Monsieur le ministre, la France n'est pas faite que de métropoles et de centres urbains qui concentreraient les actifs et les surdiplômés. Je rappelle que plus de la moitié de la population vit dans une commune de moins de 10 000 habitants. Or il se trouve que, depuis quelques années, l'État a particulièrement délaissé les habitants des territoires ruraux, qui ont le sentiment de ne plus exister, de ne plus être considérés par lui. Les manifestations de cet abandon sont multiples : fermetures régulières de services publics, recul de notre industrie, particulièrement dans les zones déjà fragilisées, disparition de commerces dans les centres-villes des petites communes, déserts médicaux et offre médicale qui reflue, et difficultés persistantes pour accéder au réseau numérique. Pourtant, les Français qui habitent dans ces territoires attendent de l'État de pouvoir bénéficier de ces services essentiels à la vie sociale et à la vie tout court. Il n'y a pas que les centres métropolitains ; je crois même que la ruralité est un acteur essentiel et qu'elle dispose d'un potentiel largement oublié dans la stratégie de l'État et dans ses politiques publiques. le sais, vous n'ignorez pas que les élus locaux de ces territoires se découragent et que même, parfois, ils désespèrent, alors qu'ils sont souvent le seul et le dernier interlocuteur public.

entre grandes agglomérations et communes rurales

La parole est à Mme Sophie Primas, pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, L'encadrement des ressources et des dépenses des collectivités, la diminution sans concertation des contrats aidés, les annulations de crédits, les engagements non respectés créent une grande inquiétude pour les élus locaux. Leur crainte est de ne plus pouvoir répondre aux demandes des populations, notamment des plus fragiles. L'autonomie financière des collectivités locales, pourtant garantie par la Constitution, est battue en brèche. La réforme hâtive de la taxe d'habitation en est une nouvelle illustration. affaiblit le pouvoir fiscal des communes et menace la pérennité de leurs ressources. Le dégrèvement est un moyen pour l'État de reprendre la main et de revenir sur la décentralisation et l'autonomie des collectivités territoriales. Cette réforme accroîtra les disparités entre communes riches et communes pauvres, elle frappera de plein fouet 20 % des Français qui acquittent déjà 80 % de l'impôt sur le revenu, elle affaiblira le lien entre le citoyen et le financement des services publics communaux. Dans 8 000 communes, on comptera moins de dix contribuables et, dans 3 000, moins de ...Voilà qui pose la question de l'acceptation de l'impôt, du respect de l'égalité devant l'impôt. Votre projet ne règle en rien les injustices qui résultent de l'obsolescence des bases locatives ; il les concentre sur quelques contribuables. Pourquoi, alors, ne pas toucher à la taxe foncière, dont les bases de calcul sont à peu près similaires ? Quel manque de cohérence et de vision ! Ne croyez-vous pas, monsieur le ministre, qu'il serait préférable, au lieu de se précipiter dans une réforme mal ficelée, de construire avec les maires et le Sénat une fiscalité moderne qui garantisse l'autonomie fiscale des collectivités et qui assure un juste lien entre le citoyen et le contribuable

secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, la suppression de la taxe d'habitation pour 80 % des foyers français a été approuvée massivement lors de l'élection présidentielle et des élections législatives qui ont suivi. Le Président de la République, à l'époque candidat à l'élection présidentielle, a mis au coeur de son projet

elle est inefficace. C'est la raison pour laquelle, dans un souci de redistribution du pouvoir d'achat, mais également au nom de l'équité fiscale entre les populations de territoires qui ne disposent pas des mêmes atouts, nous procéderons

séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2018, adopté par l'Assemblée nationale. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Bruno Retailleau. Madame la présidente,

qui fait mentir le vieux proverbe français selon lequel « tout mal guérit par la patience ». C'est bien l'impatience d'être parmi nous

le secrétaire d'État, vous pouvez compter sur le Sénat pour l'examiner sur le fond, avec cet esprit de responsabilité qui est notre marque de fabrique, sans complaisance- comptez sur nous-, mais aussi, bien entendu, sans manque

Pour être objectif, il faut pouvoir juger et apprécier un budget avec des critères. Je vous en propose deux, qui me semblent être les critères principaux. Premièrement, ce budget apporte-t-il des réponses à la hauteur de la situation de la France ? ? Deuxièmement, ce budget est-il à la hauteur de ce qu'en dit le Président de la République ? Est-ce un budget de transformation ? Pour

La dépense publique va augmenter. Certes, comme nous l'avons dit ce matin, vous n'êtes pas comptable de la dérive de la masse salariale, mais vous êtes comptable des efforts que vous pourriez faire et que vous ne faites pas,

Enfin, nous venons hier de faire l'objet de remontrances, d'un coup de semonce de la Commission européenne, qui a du mal à croire à la confirmation de vos hypothèses. Votre volonté de mettre fin à la dérive de la dépense publique, qui est un mal français,

la CSG à la TVA, qui était la seule façon de taxer les produits chinois, ... Exact ! ... d'imposer à nos frontières une sorte de régulation de la mondialisation sauvage et du social. Vous ne l'avez pas fait.

du principe du consentement à l'impôt et contredisant l'article XIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel la charge publique doit être supportée de façon équivalente et en fonction des possibilités de chacun. Ce que nous reprochons

L'année dernière, tout à votre primaire et à votre incapacité de vous mettre d'accord sur un programme présidentiel- quelles priorités ? Quel niveau d'économies : 50 milliards, 100, 120 ? Sur quelles missions ? -, vous avez, au nom d'une prétendue insincérité, préféré fuir le débat budgétaire. Rappelons que la correction des sous-budgétisations tant décriées portait, selon la commission des finances, sur environ 4 milliards d'euros,

Je sais bien, monsieur Dallier, que, quand la croissance est faible, c'est toujours à cause du Gouvernement et que, quand elle est meilleure, c'est grâce à la conjoncture. C'est toujours comme ça ! Et si l'on s'en tenait aux faits, comme nous y invite, paraît-il, le nouveau monde ?

Pour autant, nous espérons vivement que notre pays pourra enfin sortir de la procédure de déficit excessif à laquelle nous sommes soumis depuis trop d'années. Malgré la récente position de la Commission sur le déficit structurel, ce pourrait être l'une des trop rares bonnes nouvelles de ce projet de loi de finances. dernier est avant tout marqué par deux grands types de mesures : d'une part, une réduction massive de la fiscalité sur le capital, dont le coût budgétaire est malheureusement gagé par des taxes nouvelles- tabac, diesel ... -et des économies sur des politiques publiques profitant aux plus faibles, que ce soit en matière de contrats aidés ou de soutien au logement social ; d'autre part,

elle repose sur des d'inspiration libérale que nous ne partageons pas. Elle rompt tout d'abord l'égalité que nous avions instaurée en 2013 entre revenus du travail et revenus du capital, au bénéfice de ces derniers. Elle crée ensuite un biais entre investisseurs, au détriment de la pierre, et favorise par là même les plus gros revenus, ceux pour lesquels la part de l'immobilier dans le patrimoine est la plus faible.

Elle peut, de ce fait, avoir un impact sur la production de logements neufs dans notre pays. Enfin, elle sous-tend l'idée que les bénéficiaires réinvestiraient immédiatement dans l'économie productive, ce qui relève plus de la foi du charbonnier que d'une réelle expertise. La confiance de vos services est d'ailleurs telle que le retour attendu à long terme du dispositif est estimé à 0,5 point de PIB et 50 000 emplois. Par ailleurs, il est surprenant de constater, chers collègues de la majorité sénatoriale, que, partageant le même constat sur l'IFI, nous en tirions des conséquences aussi opposées. Votre volonté de supprimer totalement l'ISF se traduisant d'ailleurs par une aggravation du déficit d'environ 1 milliard d'euros que vous oubliez juste de compenser. Il aura fallu que La République En Marche ouvre la voie pour que, vous armant de courage, vous essayiez de tenir une promesse que vous n'aviez jamais jusqu'à ce jour osé concrétiser.

dont les résultats sont unanimement reconnus, voire l'Agence des participations de l'État ? En cette matière, on nous explique doctement chaque année que l'APE doit céder des parts d'entreprises pour investir dans les projets de demain ou pour conforter des fleurons nationaux.

Pour résumer, nous disons non à l'impôt sur la fortune immobilière, mais oui au rétablissement de l'impôt sur la fortune. Par pure charité, je préfère passer sous silence les différentes taxes purement cosmétiques sur les yachts et les voitures de luxe dont nos collègues de l'Assemblée nationale auraient pu se dispenser. Ça, c'est vrai ! Quand on fait des choix, on doit les assumer jusqu'au bout.

Tout d'abord, le parti socialiste a toujours considéré que cette taxe était particulièrement injuste pour les ménages et inéquitable pour les collectivités. Ensuite, il s'agit de la seule mesure qui permette de redonner rapidement un peu de pouvoir d'achat aux Français- celle consistant à prendre aux retraités pour augmenter dans le temps le salaire net des salariés n'ayant pas notre assentiment. Nous ne voterons donc pas l'amendement de suppression présenté par la majorité sénatoriale, mais nous voulons être clairs. En 2018, et les années suivantes, les collectivités locales ne doivent en rien être impactées par cette mesure de dégrèvement. Les bases nouvelles doivent être prises en compte, tout comme les éventuelles augmentations de taux. L'exposé des motifs de l'article 3, selon lequel « un mécanisme de limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par les collectivités sera discuté dans le cadre de la conférence nationale des territoires

Après moi, mon collègue Thierry Carcenac reviendra plus longuement sur l'appréciation que nous portons sur les sujets touchant plus particulièrement au financement des collectivités locales. Au moment où s'ouvre le débat sur ce projet de loi de finances pour 2018, permettez-moi de résumer ainsi la position du groupe socialiste du Sénat hostile à la réforme de l'impôt sur la fortune ; consterné par la brutalité des décisions concernant les emplois aidés et les aides au logement notamment mais ouvert à une première tranche de dégrèvement sur la taxe d'habitation, sous réserve que soit élaboré, en 2018, un projet de loi portant sur la réforme de la fiscalité locale en association avec les deux chambres. La parole

celui du logement. Je dois dire que je ne comprends pas la méthode du Gouvernement, non plus que son discours, en la matière. Chacun s'accorde à dire que nous vivons toujours une crise du logement, malgré l'embellie certaine que nous connaissons après le creux dramatique des années 2013-2015.

pourtant pas du tout ainsi que le Gouvernement aborde le problème. Certes, il affiche un discours volontariste, nous parle de réforme structurelle et de choc d'offre, mais je ne vois, dans ce PLF, que des mesures de rendement budgétaire. d'État, je ne plaide pas pour une augmentation sans fin des moyens destinés à la politique du logement, car j'ai bien conscience que les résultats ne sont pas à la hauteur des 40 milliards d'euros que nous y consacrons. Mais je ne crois pas non plus que la nécessaire réduction de la dépense publique, sans réforme structurelle préalable, sans vision d'ensemble, soit la bonne solution. Or c'est ce que vous faites dans ce PLF, à travers l'article 52, mais pas seulement. Vous supprimez

Vous supprimez la taxe d'habitation pour ne conserver que la taxe foncière, laquelle restera la variable d'ajustement des budgets communaux. Vous supprimez l'aide aux maires bâtisseurs- elle n'était pas très élevée, mais elle existait. Vous recentrez le dispositif Pinel et celui du PTZ. Vous supprimez la prime d'État pour les titulaires d'un plan d'épargne logement. Vous supprimez l'APL-accession, alors que, dans le même temps, vous souhaitez voir la vente d'HLM atteindre 40 000 logements par an- un peu de mal à comprendre votre logique. Vous taxez cette même vente d'HLM. Vous abaissez à 50 millions d'euros la participation de l'État au FNAP, rompant la promesse d'une parité entre les moyens apportés par l'État et ceux des bailleurs sociaux. Vous pérennisez le coup de rabot de 5 euros sur les APL, mesure inintelligente, selon le Président de la République, mais pérenne, puisqu'elle rapportera 400 millions d'euros en 2018. Enfin, l'article 52 de ce PLF

ce que tout le monde réclame -, vous aurez beau engager une restructuration souhaitable des bailleurs sociaux, mais qui demandera du temps pour produire des effets, vous prenez le sérieux risque de donner un coup de frein au secteur du logement.

N'avez-vous tout simplement pas mis la charrue devant les boeufs ? Il est encore temps de vous poser la question. La politique du logement est un tout, une chaîne, dont la fragilisation d'un maillon fragilisera à coup sûr l'ensemble. ce maillon faible, dans ce PLF, c'est le logement social, avec 200 bailleurs qui pourraient se retrouver au tapis dès l'an prochain. Certains seront même, dès 2018, en autofinancement négatif, et beaucoup d'autres en autofinancement si faible qu'ils auront du mal à entretenir le parc existant.

C'est oublier un peu vite, monsieur le secrétaire d'État, que tous les bailleurs ne sont pas dans la même situation : certains concentrent les publics allocataires de l'APL et seront donc particulièrement touchés par vos mesures

Vous demandez ensuite à la Caisse des dépôts et consignations de proposer aux bailleurs sociaux des prêts de haut de bilan, pour 2 milliards d'euros, considérés comme des quasi-fonds propres. Vous proposez également aux bailleurs des prêts bonifiés et un rééchelonnement prêts, monsieur le secrétaire d'État, fussent-ils bonifiés ou rallongés, restent des prêts qu'il faut un jour rembourser. Or la baisse des ressources propres des bailleurs impactera leur capacité à entretenir leur patrimoine et à construire de nouveaux logements. logements. Il n'est pas inutile de rappeler ici, au Sénat, que ce sont nos collectivités territoriales qui garantissent les prêts contractés par les bailleurs sociaux. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu d'accident- la CGLLS est faite pour cela.

de l'article 52, et même si nos collègues députés ont cherché à étaler dans le temps les effets du dispositif du Gouvernement, le compte n'y est pas. On ne peut en rester là. Le compromis que nous recherchons toujours ne peut passer que par un adoucissement de la baisse trop importante de la part de l'État pour équilibrer le FNAL.

Nous irons chercher le reste en seconde partie. Plusieurs solutions sont envisageables. Nous n'avons pas encore trouvé le bon compromis, celui qui suppose que chacun fasse de nouveau un pas vers l'autre. Le Gouvernement et les bailleurs en ont fait un premier en acceptant le principe du relèvement de la TVA.

nouvelles et baisses des dépenses, que nous pouvons encore calibrer, soit la solution pérenne sans monter en charge dans les trois prochaines années. Voilà les conditions que le Sénat y met ! Monsieur le secrétaire d'État, la balle est maintenant dans le camp du Gouvernement. Le Sénat est prêt à jouer tout son rôle. Très bien

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'effort financier consacré par l'État en 2018 aux territoires ultramarins s'élève à 17,2 milliards d'euros,

Les dépenses fiscales étant estimées à 4,2 milliards d'euros, l'effort total de l'État devrait s'élever à 21,4 milliards d'euros, selon le document de politique transversale outre-mer. Ce document présente la quasi-totalité de l'effort budgétaire et financier consacré par l'État aux territoires ultramarins. Cet effort, il faut le préciser, correspond à 3,9 % du budget général, alors que les populations ultramarines représentent 4,3 % de la population nationale, même s'il est indiqué dans le document de politique transversale que les crédits inscrits ne traduisent pas le « coût des outre-mer », mais la mise en oeuvre budgétaire des politiques publiques conduites par l'État pour ces territoires. La hausse de 1,26 % de ce budget par rapport aux exercices précédents s'inscrit dans une certaine continuité, en dépit d'une situation financière nationale toujours contrainte. Ce budget se présente comme un budget de responsabilité au regard de la priorité donnée au Gouvernement de rétablir les comptes publics de la France, transition pour les territoires ultramarins, dans la perspective des Assises des outre-mer. Le Gouvernement s'est en effet engagé à s'appuyer, pour les prochains projets de loi de finances, sur le Livre bleu outre-mer, qui résultera des Assises des outre-mer, lancées en octobre 2017

Tous les voyants sont au rouge : emploi, insécurité, immigration, éducation, finances locales, pour ne citer que ces domaines. Les maires des communes d'outre-mer que j'ai rencontrés au congrès des maires sont tous en ébullition. Les socio-professionnels sont excédés, confrontés à une chute de leurs commandes et à des grèves qui se multiplient. Tous exhortent le Gouvernement à agir urgemment,

d'État, il y a urgence à agir dès ce budget pour 2018 en envoyant des signes positifs sur des sujets très sensibles. aux accords de Guyane, qui manquent de visibilité dans ce budget, notamment le plan d'urgence qui semble avancer le frein à main tiré. Je pense aussi à la suppression brutale des contrats aidés, sujet unanime de mécontentement dans les outre-mer. des dispositions particulières pour ces territoires soient prises, mais elles mériteraient d'être davantage mises en lumière. aux dispositions d'incitation fiscale à l'investissement productif et dans le secteur du logement. Un moratoire sur la défiscalisation, en attendant d'aller plus loin, serait bienvenu.

la baisse des crédits affectés à la mobilité, à la continuité territoriale. Je pense enfin aux finances locales : la Cour des comptes a elle-même constaté, dans son dernier rapport d'octobre 2017, que le système de péréquation actuel était défavorable aux communes d'outre-mer. Sur ces différents points, je proposerai des amendements visant à offrir des opportunités de plus grande adaptation de ce budget à nos réalités ultramarines. J'espère que vous leur donnerez une suite favorable. Pour terminer, à la lumière de toutes les difficultés que vous rencontrez pour faire rentrer dans ce budget les attentes des populations ultramarines, je veux insister sur la nécessité d'instaurer dans nos territoires la la responsabilité d'un réel développement propre, de façon à sortir de cette dépendance budgétaire que vous-même vous ne souhaitez pas non plus. La croissance par les transferts publics a atteint ses limites. Le Président de la République lui-même veut donner une nouvelle marque, un nouveau souffle aux politiques publiques.

notre développement en fonction de nos réalités, de notre environnement complexe, de nos caractéristiques mentales et sociales propres. Il ne saurait y avoir d'égalité réelle sans émancipation réelle,

d'État, le « vivre ensemble », auquel vous êtes, avec le Gouvernement, très attaché, comme nous tous ici, quelles que soient nos convictions économiques, ne concerne pas seulement les individus ; il existe des structures qui le rendent possible et le font vivre,

elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » Dès lors, l'exonération des revenus des plus aisés par l'instauration, certes subtile, et néanmoins injuste, d'une « » ou par la suppression de l'ISF-

En effet, les classes dites moyennes, inférieures ou supérieures, ont le sentiment d'être les « dindons de la farce », les oubliés du nouveau monde dont vous nous rebattez tant les oreilles. Discriminer ce qui serait un investissement productif d'un autre désigné à la vindicte populaire comme improductif est également un mauvais signal adressé à nos concitoyens. C'est ainsi qu'il sera préférable d'alimenter un compte bancaire, totalement exonéré, plutôt que d'investir dans des biens immobiliers destinés à la location, opération économique qui participe de la chaîne productive et de son dynamisme. Dans nos territoires, l'adage « Quand le bâtiment va, tout va » retrouve tout son sens. Claude Raynal a déjà évoqué brillamment ces choix fiscaux inopportuns et injustes.

Pourquoi, alors que vous nous annoncez une réforme globale à venir de la fiscalité locale, procéder dans l'immédiat par ajustements, en ne menant ni travail de réflexion ni concertation approfondie avec les principaux intéressés, à savoir les représentants des collectivités locales ?

qu'en raison des valeurs locatives sur lesquelles elle est assise. Cet argument de l'injustice perdurera pour les 20 % de ménages qui resteront assujettis à cet impôt, mais également pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ce qui est injuste ici, donc, ne le serait plus là ? Qu'en est-il du devenir de l'expérimentation de révision des valeurs locatives réalisée sur cinq départements et qui a vocation à être étendue à l'ensemble du territoire national ? national ? La suppression de la taxe d'habitation, si elle s'appliquait en l'état, outre qu'elle ne résoudrait pas les problèmes d'injustice, pourrait être considérée comme

et non simplement à accroître le pouvoir d'achat. De surcroît, cette disposition mécontente et inquiète la communauté des élus. Les maires vous en ont fait part récemment au cours de leur congrès.

revenu de solidarité active, l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation du handicap et l'aide sociale à l'enfance pour les mineurs non accompagnés -, ne sont pas des dépenses de fonctionnement dont Fixer un nouveau ratio d'endettement ainsi qu'une règle d'or renforcée, qui imposerait d'affecter prioritairement les capacités d'autofinancement au désendettement, conduirait les départements à ne plus investir.

par un fonds d'urgence de 100 millions d'euros prélevés sur la CNSA, n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Le précédent gouvernement avait proposé 200 millions d'euros, et le compte n'y était pas. Je précise que certains départements ne rembourseront plus l'avance mensuelle du RSA effectuée par les caisses d'allocations familiales, décalant ainsi à l'année suivante le remboursement de cette allocation, ce qui a l'air de ne préoccuper personne, et surtout

C'est pourquoi il serait préférable d'envisager une révision générale des financements des collectivités locales, au lieu d'additionner les décisions prises en urgence, visant à sortir au coup par coup d'une impasse budgétaire

la collectivité nationale poursuit son endettement, avec une hausse de 4,5 % en 2018, qui vient d'être critiquée par la Commission européenne. L'État ne s'applique pas à lui-même la rigueur qu'il impose aux autres.

le comité des finances locales, dans le monde ancien donc, l'objectif d'évolution de la dépense locale n'avait pas de valeur contraignante pour les collectivités locales analysé en fonction de la nature des collectivités, une différenciation étant faite entre pôle communal, département et région. Qu'en sera-t-il à l'avenir ?

En macroéconomie, on évoque toujours la hausse des recettes des DMTO. Mais, là encore, en dépit d'une péréquation dite horizontale, les inégalités sont flagrantes entre les territoires.

l'examen du premier projet de loi de finances d'un quinquennat est un événement d'une grande importance pour la Nation, parce qu'il détermine d'emblée les principales orientations du Gouvernement, et ce pour cinq ans. devrait être en premier lieu l'occasion de briser un certain nombre de tabous français, s'agissant par exemple de notre addiction à la dépense publique et à une fiscalité complexe, peu lisible et, dans certains domaines, peu efficace. Il doit en outre ouvrir des pistes de réflexion pour l'avenir, en préparant des réformes difficiles mais nécessaires, qui ont été trop longtemps repoussées. Il doit enfin traduire en actes les promesses de campagne du Président de la République, afin de préserver la crédibilité de la parole publique et de concrétiser la vision politique qui a reçu l'approbation du suffrage universel. Le texte que nous allons examiner satisfait plusieurs de ces critères. Le groupe des Indépendants examinera donc de façon ouverte les orientations correspondantes de ce projet de loi de finances, mais il examinera aussi, bien entendu, l'ensemble de ce projet avec vigilance. Nous aurons également à coeur d'être force de proposition, afin d'améliorer ce projet dans le sens de valeurs qui nous paraissent essentielles : la justice sociale, la responsabilité budgétaire, une efficacité économique au service de tous et le respect d'un développement durable sur le long terme. La justice sociale, d'abord : il s'agit de faire en sorte que le travail procure les ressources qu'ils méritent à ceux qui l'exercent et que la solidarité nationale soit aux côtés des plus fragiles. est celle d'une société juste, qui donne à chacun les mêmes opportunités de réussir et ne laisse personne au bord du chemin. Nous avons porté cet objectif lors des discussions sur le PLFSS, et nous aurons la même exigence pendant la discussion du projet de loi de finances. La responsabilité budgétaire, ensuite : elle revient à faire de notre sortie de la procédure européenne pour déficit excessif une priorité. Sans ce préalable, notre politique européenne est vouée à l'échec. Malgré les efforts consentis dans le projet de loi de programmation et dans ce projet de loi de finances, le différentiel de trajectoire avec l'Allemagne est préoccupant, tant en matière de dépense publique que de désendettement. La Commission européenne a rappelé hier les interrogations qui pèsent sur l'évolution de notre effort structurel. Honorer nos engagements budgétaires et renouer avec une dépense publique saine et maîtrisée doivent être nos priorités pour l'avenir, au service d'une influence retrouvée en Europe. Sans crédibilité budgétaire, il n'y aura pas de crédibilité politique. L'efficacité économique, en troisième lieu, signifie rompre avec une logique punitive selon laquelle l'argent serait mieux utilisé par l'État que par les acteurs économiques. Il faut rendre aux entrepreneurs français la volonté d'investir dans l'innovation, dans la créativité et dans l'emploi en France. Ce projet de loi de finances contient des mesures qui vont dans ce sens, et nous ferons nous-mêmes des propositions pour restaurer la confiance des acteurs économiques et l'attractivité du territoire. défi du développement durable, c'est admettre l'existence d'une nécessité impérieuse pour notre société et pour notre planète, mais également saisir les opportunités économiques de l'avenir. Ce premier budget du quinquennat doit être l'occasion de préparer la transition de notre économie vers un modèle de production et de consommation plus responsable.

Le Gouvernement s'est employé cette semaine à rassurer les maires sur ses intentions. L'intervention du Premier ministre a permis de clarifier un certain nombre de questions. Le Président de la République s'exprime en ce moment même devant le congrès des maires, à la porte de Versailles. Néanmoins, plusieurs points demeurent encore flous ou imprécis, notamment les mécanismes de contractualisation proposés. Sans faire au Président de la République un mauvais procès sur d'éventuelles velléités recentralisatrices, notre groupe et l'ensemble de cette assemblée seront attentifs à préserver la liberté d'action des collectivités, qui agissent au plus près des Français, à leur service, au quotidien. Le groupe des Indépendants veillera à ce que les principes que j'ai évoqués soient inscrits dans ce texte et nourrissent nos débats. Nous participerons aux discussions avec un esprit constructif et nous aurons à coeur d'être force de proposition. En un mot, monsieur le secrétaire d'État, nous aurons la volonté d'agir, en responsabilité et au cas par cas, au service de l'intérêt national.

L'Europe a renoué avec une phase de croissance plus soutenue, à hauteur de 2 % environ sur l'année 2017, mais ce chiffre est encore, en France, sensiblement inférieur à la moyenne de la zone euro. notre endettement est nettement supérieur à la moyenne européenne, et ce ratio d'endettement, qui se rapproche des 100 % du PIB, ne pourra s'améliorer que très lentement au cours des prochaines années. En termes de déficit public et de balance du commerce extérieur, nous ne figurons pas non plus parmi les bons élèves de l'Europe. Ce simple constat devrait conduire ceux qui ont gouverné ou soutenu les politiques menées au cours de la dernière décennie à la plus grande modestie, ainsi qu'à une certaine réserve, dans leurs critiques et leurs propositions. Face à cette situation, notre pays doit diminuer son endettement et réduire en priorité les déficits budgétaires de l'État et des administrations sociales. Cet endettement est une véritable épée de Damoclès pesant sur nos finances publiques ; il pourrait nous plonger dans une crise budgétaire très grave si les taux d'intérêt venaient à remonter. La charge de la dette se situe déjà dans une fourchette de 40 milliards à 50 milliards d'euros par an, c'est-à-dire l'équivalent du budget de l'éducation nationale. le même temps, nous devons transformer notre économie et la rendre plus compétitive et créatrice d'emplois. En réduisant les charges sociales patronales et salariales et en allégeant la pression fiscale sur les agents économiques, nous permettrons aux entreprises de se développer par l'innovation et l'investissement. Ces mesures sont complétées par un programme de réformes sans précédent, engagées ou en préparation, qui portent sur les négociations sociales et le droit du travail, la formation professionnelle, l'apprentissage et l'indemnisation du chômage. Simultanément, nous devons conserver des leviers pour améliorer le pouvoir d'achat des Français et renforcer la solidarité à l'égard des plus défavorisés. Cette équation est difficile, mais le pari est tenable, car le Gouvernement propose une rigueur budgétaire s'appuyant sur une maîtrise des dépenses- certes, celle-ci nous paraît encore insuffisante -et non sur une majoration des prélèvements obligatoires. Cette ligne de conduite contribue au retour d'un climat de confiance avec les partenaires économiques, confiance qui est l'un des moteurs essentiels de notre attractivité, de l'investissement et du développement des entreprises. Selon un récent sondage- n'en déplaise aux grincheux -, jamais l'envie d'entreprendre dans notre pays n'aura été aussi forte et appréciée que depuis quelques mois. Ce cycle vertueux et dynamique, il nous appartient de l'accompagner, en soutenant la politique budgétaire du Gouvernement en incitant ce dernier à améliorer ses performances, tout en conservant bien entendu la liberté d'amender certaines dispositions qui ne nous paraîtraient pas adaptées aux objectifs poursuivis.

Parallèlement, il oriente les capitaux vers l'économie productive, en réformant l'ISF. Cette mesure, critiquée par des opposants de droite ou de gauche, pour des raisons d'ailleurs diamétralement opposées, remplace d'anciens dispositifs d'exonérations et de déductions fiscales complexes et peu lisibles. Si ce choix est contestable, il est assumé, et il semble quoi qu'il en soit préférable de privilégier l'activité et le travail par rapport à la rente. Pour ce qui concerne les collectivités locales, je souhaite qu'un dialogue rénové permette une meilleure compréhension. En 2018, l'enveloppe normée sera stable ; elle ne comporte donc pas de baisse de dotations. Quant à la suppression de la taxe d'habitation pour 80 % des ménages, elle sera neutre pour les collectivités assurera même une certaine liberté ou autonomie financière, dans la mesure où le taux voté donnera un produit qui sera entièrement perçu. La technique du dégrèvement est rassurante.

Concernant la maîtrise de l'évolution des dépenses des collectivités, le choix du périmètre semble judicieux ; la méthode de la contractualisation est la bonne, mais la base de négociation, c'est-à-dire l'évolution tendancielle des dépenses de fonctionnement, n'est pas acceptable.

Nos craintes portent également sur la politique du logement, qui, si elle n'est pas amendée, pourrait avoir des effets contraires aux objectifs poursuivis : le risque est d'accentuer les fractures territoriales au détriment des régions et des territoires les moins attractifs. Il conviendrait,, d'améliorer l'atterrissage du dispositif Pinel et d'aborder avec plus de discernement le financement de la baisse des APL. Si certains opérateurs sociaux disposent de réserves significatives, d'autres risquent d'être fragilisés par l'assèchement de leurs capacités d'autofinancement et seront conduits à renoncer au lancement de nouveaux programmes.

: sortir des errements du passé et favoriser la réussite de la France. Sachez, monsieur le secrétaire d'État, que vous trouverez chez nous une volonté de participer à la réalisation de cette ambition, même si nous n'en partageons pas toutes les modalités. Ce projet de loi de finances s'inscrit dans un contexte assez particulier, qu'il convient de rappeler : faible inflation, taux d'intérêt toujours extrêmement bas, bas, matières premières bon marché, embellie économique de la zone euro, avec, en France, une croissance sensiblement plus élevée qu'au cours des dernières années,

déficit important et préoccupant de notre commerce extérieur et, surtout, très fort niveau d'endettement, aujourd'hui à la limite du soutenable.

du fait que le Sénat représente les collectivités locales pour ne pas opposer deux légitimités démocratiques récentes : celle des élus locaux, les maires, élus préférés des Français ; et celle du Président de la République, dont la légitimité est toute fraîche. Faisons en sorte de concilier ces deux légitimités

pour défricher utilement des voies nouvelles permettant à notre pays de retrouver une place plus conforme à ses ambitions, grâce à une situation économique, financière et sociale devant nous placer en tête du peloton européen. Ainsi, nous répondrons à l'objectif

les mesures prises par le Gouvernement à l'égard de l'AEFE, en coupant les subventions de 33 millions d'euros, vont porter une grave atteinte à notre réseau d'enseignement français à l'étranger, alors que le ministère de l'éducation nationale bénéficie pour la France d'une hausse de 1,3 milliard d'euros.

Le Président de la République s'était engagé devant les élus de l'AFE à ne pas diminuer les crédits en 2018 et en 2019 : « Les crédits de l'AEFE seront préservés à partir de 2018, ce qui veut dire, à mes yeux, pour les deux années consécutives, parce qu'il faut de la visibilité pour développer une stratégie et parce que le défi est un défi tant en termes de crédit que parfois en termes de réorientation qualitative du réseau et on ne peut pas de manière crédible, comme je l'ai fait et comme je le crois profondément, dire qu'on est pour que la France à l'étranger accompagne celles et ceux qui vivent et que vous représentez et dire que, l'un des enjeux fondamentaux de notre bataille, c'est la francophonie et ne pas s'en donner les moyens. Le Président de la République avait été très applaudi. Malheureusement, en 2017, c'est 33 millions d'euros de crédits qui venaient d'être supprimés sans préavis, sans que les élus en aient pris conscience. Une décision prise fin novembre pour une application début janvier est clairement impossible. Les établissements conventionnés ne sont pas des centres de profit. Leurs budgets sont gérés au plus juste pour limiter les charges sur les familles vivant à l'étranger. Un changement de cotisation en cours d'année scolaire signifie une augmentation des tarifs non provisionnée par les familles. Même dans le cas d'un report à la rentrée de septembre, bon nombre de lycées français à l'étranger feront le choix de modifier leur partenariat avec l'AEFE. En commençant par le déconventionnement, certains lycées pourraient être tentés d'aller plus loin par manque de confiance à l'égard de leur partenaire. Ce serait une perte d'influence pour la France, puisque beaucoup d'établissements scolaires français de l'étranger sont également fréquentés par des enfants venant de la population locale pour eux, c'est un enseignement d'excellence. Au contraire d'une diminution, nous devions obtenir des crédits supplémentaires pour que les parents d'enfants avec des besoins particuliers puissent bénéficier d'une aide pour payer les assistantes de vie scolaire qui les accompagnent. d'un dépistage précoce leur permettant d'être pris en charge le plus rapidement possible, leur donnant ainsi une véritable opportunité de réintégrer notre système. Au lieu de cela, nous continuerons à avoir des enfants déscolarisés, qui restent à la maison, faute d'être pris en charge dans les établissements scolaires français à l'étranger, et qui seront à la charge de leurs parents et de la société jusqu'à la fin de leurs jours.

L'examen du projet de loi de finances et de ses nombreuses missions a mis en évidence le travail de grande qualité des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis, ainsi que celui de l'ensemble du personnel de la Haute Assemblée. un objectif extrêmement complexe pour un gouvernement, quel qu'il soit. En effet, le déficit budgétaire se dégrade pour atteindre en 2018 près de 83 milliards d'euros. Dans le cadre de l'examen de la mission « Engagements financiers de l'État la charge de la dette s'élève à 40,24 milliards d'euros, soit l'un des postes budgétaires les plus importants. L'encours de la dette a progressé de 17 % de 2012 à 2016 et progresse de 4,5 entre 2017 et 2018 pour atteindre un montant exceptionnel de 1 752 milliards d'euros. La situation est très grave. Comment respecter l'engagement européen de maintenir le déficit

Il est incontestablement nécessaire, cela a été rappelé par de nombreux collègues, de donner la priorité au développement économique et au monde des entreprises. S'agissant des dépenses totales, elles s'élèveraient en 2018 à environ 441 milliards d'euros tout confondu. Comment maîtriser les dépenses ? La tâche reste immense depuis de nombreuses années, alors que nous devons faire face à des enjeux importants. Certaines missions doivent être renforcées : le budget des armées, la sécurité intérieure,

En outre, j'aborderai le partenariat indispensable- et de confiance -entre l'État et les collectivités territoriales. Plus de 40 milliards d'euros sont prélevés sur les recettes de l'État pour aider au financement des collectivités territoriales. L'État est donc le premier partenaire financier des sont particulièrement inquiets concernant les dotations de fonctionnement ; je pense en particulier à la DGF, ce qui a été maintes fois évoqué. L'autonomie financière des communes et des intercommunalités avec la suppression à court terme de la taxe d'habitation. S'agissant de l'investissement des collectivités locales, domaine important pour la relance du bâtiment et des travaux publics, des incertitudes subsistent sur les répartitions de la DETR, du FSIL, sans oublier la disparition de la dotation d'action parlementaire- ex-réserve parlementaire -, soit une perte de plus de 140 millions d'euros à destination en particulier

Le Gouvernement assurera ce débat avec le sens aigu des responsabilités qui lui incombe en ce moment particulier que traverse notre pays, avec la plus grande des sincérités et avec la certitude qu'ici, au Sénat,

la vie quotidienne, de la mobilité, de l'accès au très haut débit. Je reviens de Normandie, et j'en ai dit un mot tout à l'heure lors des questions d'actualité au Gouvernement. Bref, c'est un pacte global qui ne se limite pas simplement à la question du montant du pouvoir d'achat.

un gain d'un peu plus de 850 euros par an à la fin du quinquennat. Ce gain de pouvoir d'achat est particulièrement renforcé pour nos compatriotes qui ont les revenus les plus fragiles.

les grandes institutions bancaires et avec nos partenaires à la mise en place de nouveaux produits permettant d'orienter l'épargne des Français vers l'appareil productif, vers l'investissement et vers nos entreprises. Je ne reviendrai pas trop longuement sur la taxe d'habitation, car je suis certain que nous aurons l'occasion d'en débattre dans les jours et les semaines qui viennent.

collectivités locales. Mais le débat lors de l'élection présidentielle a été fort sur la question de la réduction des dépenses publiques. Le Président de la République s'était engagé sur une baisse de 13 milliards

Le principe qui est le nôtre, dans le dialogue exigeant que nous allons engager avec les collectivités, est celui de la responsabilité partagée. Nous voulons finalement donner aux collectivités locales la liberté secteurs où elles souhaiteront faire porter l'effort. L'un d'entre vous a cité François Mitterrand. Je suis petit-fils de Morvandiau, d'Autun, pas très loin de Château-Chinon où le Président de la République élu le 10 mai 1981 au soir a réuni les élus locaux dont il avait été président de conseil général pendant de nombreuses années. Sa première phrase a été de leur dire, lui qui aimait les mots : « Ce pouvoir que les Français m'ont confié, je vais vous le rendre ! C'est dans cet état d'esprit que nous travaillons, comme l'a rappelé le Président de la République cet après-midi dans son intervention : un esprit de liberté et de responsabilité partagé entre l'État et les collectivités locales. C'est un ancien élu départemental qui vous le dit.

C'est une décision qui permet de donner de la lisibilité, de la visibilité et de la transparence à beaucoup de responsables et de chefs d'entreprise.

l'économie de la connaissance, de la compétence et de l'innovation. C'est le crédit d'impôt recherche sanctuarisé pour nos entreprises, c'est la création du fonds pour l'innovation de rupture, financé à hauteur de 10 milliards d'euros par les cessions de participations dans des entreprises publiques, que nous assumons parfaitement.

de me déplacer à l'étranger dans le cadre des différentes missions qui m'ont été confiées. Le fait que l'Autorité bancaire européenne déplace son siège à Paris, le fait que quelques grandes banques et quelques grands fonds aient fait le choix de se relocaliser à Paris après les procédures engagées dans le cadre du Brexit sont des premiers signaux.

dans la réforme qui a été engagée sur le marché du travail, est de réconcilier enfin le capital et le travail dans notre pays. Je suis certain que nous pouvons y arriver. À n'avoir fait le choix que de l'un ou de l'autre, alternativement, nous avons réussi le miracle de n'avoir aucun des deux : nous manquons de financement pour nos entreprises et nous avons

la question du logement social. Je ne doute pas que l'article 52 du projet de loi de finances sera abondamment discuté. Je ne voudrais donc pas priver les gourmands

travailler à avancer sur tous ces sujets. L'Assemblée nationale a adopté le principe de détendre les dispositifs qui devaient, pour certains d'entre eux, s'arrêter de manière brutale le 31 décembre de cette année.

L'article liminaire que nous nous apprêtons à voter est important ; il fixe en effet la prévision de soldes structurel et effectif de l'ensemble des administrations publiques. Dit autrement, il pose le cadre du débat parlementaire sur le projet loi de finances. Le groupe La République En Marche est très fier de défendre ce budget, qui, comme l'a noté le rapporteur général, dont je salue le retour parmi nous, est un budget de sincérité.

Or, vous le savez, cette réévaluation rend l'effort à mener par le Gouvernement plus important. Le rapporteur général l'a aussi noté, le texte que le Sénat examine est un texte de responsabilité.

pays dont la dépense représente 56 % du PIB, va enfin opérer une baisse dans ce domaine. Oui, c'en est fini des hausses d'impôts pour éviter de transformer le pays et de faire les réformes Cette responsabilité permet à la France de passer durablement sous le seuil de 3 %. Il y a eu beaucoup à faire en 2017, par exemple trouver 10 milliards d'euros à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de la taxe à 3 % sur les dividendes, mais la majorité présidentielle a tenu son cap. À cet égard, notre groupe regrette une nouvelle fois le

très lourdes baisses de dépenses publiques. Elles seront subies, une fois de plus, par ceux qui ont pour seul capital le service public. Vous évoquez la société du risque ; il est sûr que les Français les plus modestes vont en subir les effets.

Il nous a répondu que « les problèmes de soldes structurels ont fait l'objet de travaux qui n'ont pas été validés par les ministres des finances ». Il est vrai que nous n'avons pas entendu le Gouvernement sur ce dossier, pourtant essentiel pour respecter nos engagements européens, tout en préservant nos services publics et en répondant à l'urgence sociale. cela, préserver nos services publics et répondre à l'urgence sociale, ne semble pas être votre problème. À quoi sert un gouvernement de la zone euro si les règles actuelles étranglent l'action publique de l'État, vecteur majeur de redistribution ? le voit bien, même les meilleurs élèves de l'Europe subissent des crises politiques liées aux montées des nationalismes, lesquels sont exacerbés par la hausse des inégalités. Parce que la vertu d'un pays européen n'est pas mesurée par sa situation sociale, mais par un calcul baroque de solde structurel, dont tout le monde sait qu'il n'est que très théorique. Pour conclure, vous avez utilisé les marges de manoeuvre existant sur cet exercice pour favoriser les plus aisés au détriment des plus défavorisés, sans satisfaire pour autant la Commission vous n'avez pas renégocié le mode de calcul de ce fameux solde structurel ; vous n'avez pas cherché, et vous ne chercherez pas, à utiliser les flexibilités prévues par le TSCG, notamment la non-prise en compte dans le déficit des dépenses de défense. Vous opposerez certainement à mes arguments vous parlez d'addiction à la dépense publique. Je pense surtout que notre société a une addiction à la pauvreté et au creusement des inégalités, ce dont, finalement, vous vous satisfaites.

après l'invalidation par le Conseil constitutionnel de la taxe sur les dividendes, laquelle entraîne une perte de 10 milliards d'euros pour l'État en 2017-2018. Comme on l'a vu lors des débats prolongés du premier projet

Comment informer nos concitoyens, comment les mobiliser sur la nécessité de redresser nos finances si on ne leur parle pas dans la monnaie de leurs propres comptes ? L'article liminaire a été imposé par la loi de 2012 pour donner une image fidèle et synthétique de l'évolution de nos finances. Tel que rédigé, il est incompréhensible pour le commun des mortels.

du montant de la contribution de la France au budget européen pour l'année 2018. Le vote de cet article, même s'il est contraint, est l'occasion pour le Parlement d'apprécier chaque année la pertinence des priorités européennes mises en oeuvre. L'année 2018 s'inscrit dans un contexte particulier : le Brexit et les négociations en vue de son dénouement, l'arrivée à mi-parcours de la programmation 2014-2020, le contexte lié à la prénégociation du programme de l'après-2020. Pour rappel, la France se plaçait en 2016 à la deuxième place des contributeurs nets en volume, après l'Allemagne. Notre pays était, dans le même temps, le troisième bénéficiaire en volume des dépenses européennes, après l'Espagne et l'Italie. Ce budget de l'Union européenne bénéficie de manière très concrète à l'ensemble de nos territoires, ce qui n'est pas toujours correctement perçu par la population française, qui témoigne, comme la population d'autres pays européens, d'une certaine défiance à l'égard de l'Union. l'égard de l'Union. Je pense bien entendu à la politique agricole commune, qui contribue à garantir un revenu aux agriculteurs, concourt à l'aménagement de notre territoire et accompagne les efforts des agriculteurs vers la transition écologique. J'aurais pu également citer le Fonds européen pour les investissements stratégiques mis en place dans le cadre du plan Juncker, qui permet aujourd'hui de soutenir 57 projets sur l'ensemble du territoire, et dont la France est l'un des premiers bénéficiaires. L'article 27 du projet de loi de finances pour 2018 évalue le montant de la contribution française à 20,2 milliards d'euros, soit une hausse de 3,8 milliards d'euros par rapport au montant qui devrait être effectivement payé en 2017. Cette progression s'explique essentiellement par la montée en charge des programmes de la politique de cohésion, après plusieurs années de sous exécution en début de programmation. Le 18 novembre dernier, le Conseil et le Parlement européens sont parvenus à un accord sur le budget, pour un montant légèrement inférieur à celui proposé par la Commission européenne. Madame la ministre, dans la mesure où les crédits proposés dans le projet de loi de finances étaient fondés sur les chiffres de la Commission, le montant du prélèvement le montant du prélèvement sur les recettes pour 2018 fera-t-il l'objet d'un ajustement à la baisse, comme cela était le cas pour les crédits prévus initialement au titre de l'année 2017 ? 2018 verra s'intensifier les négociations en vue de la programmation pour l'après-2020. À cet égard, un certain nombre de défis se posent à l'Union : comment combler la perte nette de recettes consécutive à la sortie du Royaume-Uni ? Comment financer de nouvelles priorités- la transition écologique, les enjeux migratoires ou la lutte contre le chômage des jeunes -sans sacrifier la politique agricole commune et la politique de cohésion ? Comment rééquilibrer le système de ressources propres ? Depuis les années 1980, le budget européen dépend principalement des contributions des États membres. Or les budgets nationaux sont de plus en plus sous pression. Les États tentent de limiter leurs contributions au financement de l'Union, afin de réduire ce qu'ils considèrent comme un coût sur le budget national. C'est pourquoi il est urgent que l'Europe se dote de ressources propres. Cette réforme du système des ressources propres doit être l'occasion de faire avancer l'harmonisation fiscale en Europe et de lutter contre la concurrence déloyale entre États membres qui, le scandale des « Paradise papers » nous Parmi les pistes en cours de discussion, le projet d'harmonisation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés est certainement le plus ambitieux. Fondé sur le principe selon lequel « les impôts sont payés là où les bénéfices sont réalisés », il présenterait l'avantage d'accroître la justice fiscale, tandis qu'une part de son produit pourrait être affectée au budget de l'Union. Des options plus pragmatiques, comme une taxe sur les chiffres d'affaires des grandes entreprises du numérique, les fameux GAFAM, doivent et peuvent être adoptées rapidement. Sur ces sujets, il importe en effet de progresser vite, car les attentes de nos concitoyens sont fortes. C'est une question de justice fiscale et sociale. S'agissant des conséquences du Brexit, qui entraînera une perte de recettes d'environ 10 milliards d'euros nets par an, il nous faudra être vigilant sur la politique de cohésion. En effet, pour équilibrer le budget de l'Union, plusieurs pistes de réduction des dépenses sont à l'étude. Parmi elles, une baisse de 15 % à 30 % des crédits affectés à cette politique. Cette politique est d'autant plus fragilisée que d'importants retards de mise en oeuvre sont constatés dans tous les États membres, dont la France. La lourdeur des procédures de contrôle et d'audit semble y être pour beaucoup, mais aussi la prolongation du délai de mise en oeuvre du dégagement d'office. Cette situation est dommageable pour les porteurs de projet, mais elle fait aussi peser un risque sur la bonne exécution du cadre financier. Pourtant, la politique de cohésion constitue un lien essentiel entre l'Union européenne et les collectivités territoriales, y compris les plus pauvres et les plus isolées. À cet égard, la prise en compte de territoires homogènes au regard de leur richesse dans le cadre de la nomenclature des unités territoriales territoriales statistiques constitue un enjeu essentiel pour l'avenir. Permettez-moi enfin d'insister sur le fait que le budget européen que nous voulons pour demain doit nous permettre de renforcer la vocation d'origine de l'Union, qui est d'assurer la prospérité, la solidarité et la lutte contre les inégalités. Il nous faut aussi donner à l'Union les moyens nécessaires pour être une puissance d'avenir, à la fois compétitive et capable de faire évoluer son modèle de développement. C'est à cette condition que l'on renforcera la souveraineté européenne garantissant la démocratie, la liberté et la paix. En conclusion, pour revenir sur le seul aspect budgétaire, je recommande, au nom de la commission des finances, l'adoption sans modification de l'article 27 du projet de loi de finances pour 2018. La parole

Après lui, je constate la progression de la contribution de la France. Cette évolution doit nous conduire à prendre conscience des trois défis que le budget européen est appelé à relever, avec les conséquences qui en résultent pour la contribution de notre pays. Le premier défi regroupe les nouvelles priorités que l'Union européenne est appelée à assumer, avec leurs conséquences budgétaires : la sécurité, le contrôle des frontières, le terrorisme, la défense, les crises migratoires-autant de défis et d'attentes qui sont également ceux de nos concitoyens. Le deuxième défi est d'avoir un budget européen adaptable à l'imprévu, sinon à l'imprévisible. La crise migratoire a démontré la difficulté pour l'Union de trouver rapidement, dans ses procédures budgétaires, la flexibilité nécessaire à des réponses efficaces. troisième défi est la réduction programmée des ressources budgétaires de l'Union. Le Brexit, tout comme la nécessaire maîtrise des budgets nationaux, va peser sur la marge d'action financière des politiques européennes. Pour bon nombre d'États membres, dont la France, le Brexit entraînera, à budget européen constant, une contribution plus élevée au budget européen. Ces trois défis doivent conduire à réinventer le cadre budgétaire sous au moins trois aspects. Premièrement, il faut avancer sur la question des ressources propres, qui sont aujourd'hui insuffisantes, autour de 25 % à 28 %. Il est nécessaire que la contribution des États au budget de l'Union européenne ne soit plus, comme le rappelait M. Monti, un simple enjeu de « juste retour ». Des propositions précises sont désormais sur la table des gouvernements, qui doivent s'en emparer. Deuxièmement, le moment est venu d'établir des priorités et de les hiérarchiser. À cet égard, un critère doit prévaloir, celui de la valeur ajoutée européenne. C'est à l'aune de ce concept que seront désormais mesurées la légitimité et l'acceptation politiques européennes. Troisièmement, deux politiques sont en particulier concernées : la politique agricole commune et la politique de cohésion. L'exercice de réflexion est bien sûr nécessaire, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. La PAC, c'est un mécanisme de gestion des marchés, qui permet de prévenir les crises et d'assurer la protection de la partie vulnérable des populations agricoles européennes. C'est aussi un enjeu essentiel de sécurité alimentaire, de développement durable, de climat et d'environnement. La politique agricole relève donc, à mon sens,

Mais nous avons besoin d'un véritable « choc » de simplification administrative et de mise en cohérence des fonds. Il est bien évident que, dans une période de contrainte budgétaire nationale, ces fonds de cohésion ont aussi, à l'adresse des maires de notre pays, une lisibilité plus forte encore. Ils visent les mêmes cibles, mais avec aujourd'hui des réglementations concurrentes, sinon contradictoires. Il faut rationaliser les règles complexes de contrôle et d'audit qui bloquent cette politique

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, La France est solidaire de l'Europe, quoi qu'elle fasse et quoi qu'elle veuille. Elle l'a été dans la souffrance, elle l'est dans son économie, elle le sera dans son destin. La France a une tâche européenne qu'elle ne peut éluder ». Je sais qu'il est de bon ton de citer Albert Camus, même si

de l'Europe, ont été écrits au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans une Europe exsangue qui venait de se déchirer comme jamais auparavant. Ils méritent, à mon sens, d'être rappelés aujourd'hui, à une époque où notre continent est traversé par de multiples crises et s'interroge sur son avenir, sa cohésion et le sens à donner encore aux mots de solidarité entre les peuples et les nations qui le composent. Ces superbes mots de Camus ne sont sans doute pas si incongrus et inutiles

article : quelle Europe voulons-nous et de quels moyens sommes-nous prêts à nous doter pour y parvenir ? Mais, avant d'effleurer cette question, je voudrais procéder à un ou deux constats, qui résultent de la lecture strictement comptable comptable de cet article. Premier constat : la contribution de la France au budget de l'Union européenne augmente de 8 % par rapport à l'an passé, après avoir connu une baisse par rapport à l'exercice antérieur. Je m'en réjouis fortement, car, même s'il ne s'agit que de l'une des variables qui impactent le calcul de notre niveau de contribution, cela signifie que notre revenu national brut s'améliore et surtout que les données prévisionnelles de la Commission européenne qui fondent ce calcul témoignent d'une confiance retrouvée en notre économie, en tout cas en la sincérité de nos comptes. Second constat : la France est, après l'Allemagne, le deuxième pays contributeur au budget de l'Union. Mais ce que ce

bénéficiaire en volume des aides accordées par l'Union. Certes, et très formellement, la France reste un contributeur net d'environ 9 milliards d'euros. C'est le sens même de la solidarité entre nations et régions sur laquelle s'est fondée, puis a prospéré, l'Union européenne depuis sa création. C'est cette solidarité qui a aussi permis d'instaurer une paix durable au sein de l'Union, et il est bon aujourd'hui, je crois, de le rappeler. En réponse à celles et ceux qui, à gauche comme à droite- surtout à l'Assemblée nationale, dont j'ai relu les travaux portant sur cet article -, entament aujourd'hui l'antienne thatchérienne du « », il est bon aussi de rappeler que cette contribution nette de la France, qui les gêne tant, n'intègre naturellement pas les apports positifs du plan Juncker en matière d'investissements dans notre pays et moins encore la dynamique positive- évidente, mais plus difficile à chiffrer précisément -pour notre économie de notre appartenance à l'Union. Ceux qui doutent encore de cette dynamique n'ont qu'à se pencher sur ce qui commence à se passer de l'autre côté de la Manche depuis la décision de nos voisins britanniques de quitter l'Union. Madame la ministre, précisément parce que la nature de la construction de notre budget national laisse à penser que l'Europe nous coûte beaucoup plus cher qu'elle nous rapporte, j'avais il y a quatre ans, dans un rapport sur la citoyenneté européenne

produise annuellement un rapport largement publicisé qui évalue plus formellement les apports concrets de l'Europe à l'économie de notre pays. Le gouvernement de l'époque, en dépit du soutien de mon ancien président de commission Simon Sutour, n'a jamais donné suite à cette suggestion, car il considérait sans doute

et dans le reste de l'Union une large consultation de nos concitoyens sur notre avenir commun, je crois qu'il serait bon d'envisager à nouveau l'opportunité d'une telle publication, bien plus pédagogique que les chiffres que nous étudions ici. Pour conclure mon propos, je veux souligner ici combien la question du budget de l'Union est capitale et dépasse largement le strict enjeu financier.

cadre pluriannuel financier de l'Union, ayons le courage de tirer les conclusions du cadre financier 2014-2020, qui touche bientôt à sa fin. Le malthusianisme qui avait présidé à sa construction finale nous a profondément handicapés, nous contraignant à des logiques excessives de fongibilité entre les différents chapitres de ce cadre

tout le monde s'accorde à penser qu'il est aberrant de bâtir un cadre financier pour sept ans, surtout quand celui-ci dépend presque exclusivement des contributions nationales des États membres et n'offre aucune véritable marge de manoeuvre en cours de route. Veuillez conclure,

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, notre débat sur la participation de la France au budget de l'Union européenne intervient en un moment très particulier. En effet, dans un rapport publié le 16 novembre dernier, la Cour des comptes européenne dressait un bilan accablant des trois plans européens prétendument destinés à « aider » la Grèce. Dans le même temps, nous apprenions que la Banque centrale européenne avait réalisé 7,8 milliards d'euros de plus-values entre 2012 et 2016 sur ses rachats de titres grecs et qu'elles seraient redistribuées aux banques centrales nationales de la zone euro. Ainsi, le budget dont nous discutons aujourd'hui est nourri des misères imposées au peuple grec, de la même façon que Kronos, « le dieu aux pensées fourbes », dévorait ses enfants pour assurer son pouvoir. Après sept années de gestion directe de la Grèce par la troïka, ce pays est exsangue. La politique dogmatique et implacable de la Commission européenne a consisté à réduire drastiquement les dépenses publiques et à augmenter sans fin, dans les mêmes proportions, la la pression fiscale. Cette saignée a eu les mêmes résultats que les purges imposées par le pseudo-médecin Diafoirus de Molière à ses patients, qui mouraient guéris. Après cette cure dévastatrice, la Cour des comptes européenne constate que la pauvreté de la Grèce est terrible, que les jeunes actifs ont quitté le pays, que l'économie est toujours aussi atone, que le système financier est totalement délabré et que la dette est à un niveau tellement insoutenable qu'il est douteux qu'elle puisse être remboursée un jour. La même Cour considère que les politiques économiques appliquées à la Grèce étaient totalement inappropriées et conclut son bilan par ce constat : « En l'absence de feuille de route stratégique pour stimuler les moteurs potentiels de la croissance, la stratégie d'assainissement budgétaire n'a pas été propice à la croissance. » Gardons à l'esprit cette appréciation, nous qui allons voter, pour notre pays, un budget dont l'esprit est très proche de celui qui a été imposé à la Grèce. Il est à craindre en effet que l'austérité sévère que vous imposez à la dépense publique et la ponction fiscale supplémentaire dont vous affligez les foyers qui gagnent le moins aient des conséquences désastreuses sur la consommation. Ces efforts supplémentaires ont été jugés insuffisants par la Commission européenne, qui considère que le déficit structurel de la France va continuer de s'accroître dans des proportions qu'elle estime à 0,4 point de PIB. Sur cette pente et dans la logique de l'ordolibéralisme, les efforts ne vont jamais assez loin. Des organismes internationaux, comme le FMI et l'OCDE, recommandent l'abandon de cette politique de l'offre pour engager une politique volontaire de soutien de la demande. Pourquoi ne sont-ils pas entendus par la Commission européenne et le Gouvernement ? Le Portugal a eu le courage politique de sortir des ornières dans lesquelles on voulait le maintenir en augmentant le salaire minimum de 15 %, en réduisant le temps de travail des fonctionnaires, en bloquant les privatisations et en relançant des grands projets d'aménagement. Ces mesures l'ont engagé dans un cercle vertueux de croissance qui le place aujourd'hui dans une situation sociale et économique bien meilleure que celle de la France et qui lui permet même de respecter les critères de la Commission européenne avec un déficit public ramené à 1 % en 2018. Une autre politique budgétaire est donc possible ! La France, parce qu'elle est l'un des principaux contributeurs au budget de l'Union européenne, dont elle apporte 15 % du montant total, et parce qu'elle verse 5 milliards d'euros en sus de ce qu'elle reçoit, aurait toute légitimité pour demander à la fois un bilan critique des politiques économiques coercitives mises en oeuvre par la Commission et un examen poussé de l'efficacité du budget de l'Union européenne ainsi que de la pertinence des actions entreprises. En effet, il y a urgence à renouer le lien social entre l'Europe, ses citoyennes et ses citoyens. L'essor continu et général des partis d'extrême droite racistes et xénophobes, y compris en Allemagne, et les mesures ouvertement contraires aux valeurs humanistes européennes par lesquelles plusieurs États de l'Union y répondent sont autant de symptômes de la crise sérieuse traversée par l'Europe. Elle est de moins en moins perçue comme l'horizon d'attente d'une construction politique au service de la paix et de l'émancipation humaine et de plus en plus comme un empilement de structures bureaucratiques à la disposition d'un pouvoir économique qui agit contre l'intérêt des peuples. Nous avons besoin d'une nouvelle Europe qui les protège et les aide dans leurs projets d'émancipation, une Europe qui encourage la constitution d'une communauté fondée sur le partage de nos valeurs communes. La froide rigueur comptable de cet article 27 ne contient rien de tout cela. Nous voterons contre. La

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'Europe a été « trop faible, trop bureaucrate, incapable de répondre aux enjeux qui se présentaient à elle ». Combien de fois avons-nous entendu ces critiques critiques souvent fondées ? Aujourd'hui, pourtant, j'ai le sentiment que les discours évoluent. Malgré, ou peut-être grâce, au Brexit, l'Europe redevient porteuse d'espoir. « L'avenir de l'Europe est bien plus important que le Brexit », disait voilà quelques jours Angela Merkel. Confrontés au risque de voir exploser ce modèle de société construit depuis quarante ans, nous mesurons les choix qui se présentent désormais à nous. Voulons-nous moins d'Europe, comme le Royaume-Uni- et, si oui, pour évoluer vers quel modèle de société ? -, ou voulons-nous une Europe solidaire et renouvelée renouvelée dans son organisation, dans sa méthode, dans ses missions, une Europe apte à relever les défis ? Nombreux sont ceux qui partagent la vision ambitieuse du Président de la République, prônant une Europe de la confiance, de la convergence, qui s'empare des sujets stratégiques et, comme le disait Jean-Claude Juncker, « s'occupe davantage des grands sujets et moins des petites choses ». Cette recherche d'efficacité oblige à de grands pas en avant en matière de création d'un budget propre à la zone euro, d'un ministère des finances, d'une Europe de la défense, de lutte contre le terrorisme avec un parquet européen, de politique migratoire avec un office européen de l'asile pour harmoniser les procédures, procédures, de police aux frontières, de lutte contre le social, de taxation des géants du net, de transition écologique ou encore d'aide au développement. L'Europe doit devenir audacieuse, oser « avancer » plus vite et plus loin, quitte à organiser plusieurs niveaux d'intégration, favorisant les « avant-gardistes » sans pour autant exclure les moins intrépides ; une Europe unie- mais pas uniforme uniforme -, démocratique et souveraine, qui se numérise et innove dans le cadre d'un marché unique alliant protection, exigences sociales, environnementales et stratégie commerciale. La France et l'Allemagne ont un rôle moteur à jouer pour fonder cette nouvelle Europe. Le rapport des commissions des affaires européennes et des affaires étrangères du Sénat sur la relance de l'Europe propose une série de mesures propices à renforcer la légitimité démocratique dont a tant besoin l'Union européenne pour renouer la confiance nécessaire. Il préconise l'association et la reconnaissance des parlements nationaux, voire des citoyens, pour lancer des initiatives, interpeller les représentants et engager des débats. La reconstruction reconstruction doit partir des peuples pour insuffler l'envie d'Europe. Aujourd'hui simples gardiens du principe de subsidiarité, les parlements nationaux pourraient, demain, déléguer à une convention restreinte, chargée de statuer souverainement à la majorité qualifiée sur les mesures économiques et financières, notamment lorsqu'elles impliquent une modification du traité fondateur. Quant à la Commission, elle doit devenir le véritable gouvernement européen, responsable devant son parlement. Ainsi, les citoyens européens pourraient identifier clairement et, s'ils le jugent opportun, renverser ceux qui détiennent les responsabilités. Il est inacceptable pour les salariés, les entreprises et les gouvernants que des conditions de travail et de protection sociale déséquilibrées puissent subsister, comme cela a été le cas avec la directive dite « Travailleurs détachés ». L'initiative de la France de la réviser est déterminante pour la cohésion à venir de l'Europe. La convergence fiscale doit s'imposer, pour limiter le entre les différents États membres. Elle nous permettra également de nous protéger des stratégies d'optimisation de certaines multinationales, dont les GAFA sont les exemples les plus frappants. Une Europe qui adopte des règles justes et équilibrées, qui ne s'imposent pas au détriment des citoyens ou des acteurs économiques, que ce soit à l'échelle du marché unique, mais aussi dans le cadre des traités internationaux, internationaux, c'est le préalable d'une Europe puissante et convergente. Cette Europe sera propice aux initiatives, au développement économique, à l'innovation technologique, à une véritable politique économique commune servie par l'intégration budgétaire et une fiscalité propre. Le gouvernement économique de la zone euro, doté d'une légitimité politique, sera l'interlocuteur de la Banque centrale européenne en matière de stratégie monétaire. Il sera compétent pour adopter des politiques industrielles communes, dans des domaines clés et stratégiques, tels que le numérique, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, la transition énergétique, l'aérospatiale, afin d'additionner les atouts de nos secteurs d'activité les plus performants, d'assurer les nécessaires transitions tout en réduisant les coûts, et aussi de garantir nos approvisionnements et notre indépendance technologique. Dans cette nouvelle donne stratégique, une nouvelle politique agricole commune a toute son importance, même si, avec le temps, l'actuelle PAC s'est diluée dans autant de politiques nationales, perdant ainsi sa capacité à incarner un dessein européen. La PAC mobilise aujourd'hui 43 % du budget européen, dont 17 % reviennent à la France. Face aux perspectives, il y a lieu de s'interroger sur les conditions de sa subsistance. Pourtant, l'enjeu alimentaire du XXI siècle est incontournable, mais pas seulement. Nous avons plus que jamais besoin d'une politique agricole commune à l'échelle européenne pour assurer à nos concitoyens une alimentation de qualité et en quantité, dans une logique de développement durable, et pour relever le défi de l'évolution climatique, de la préservation des ressources naturelles et des énergies renouvelables. En ce sens, les agriculteurs européens doivent s'approprier ces enjeux et développer des outils technologiques innovants au service d'une agriculture alliant performances économiques et environnementales. Pour atteindre ces objectifs, la question du montant du budget européen, pilier d'une relance de l'Union européenne, est donc centrale. Pour nous, centristes, la participation de la France, à hauteur de 20,2 milliards d'euros Nous sommes tous conscients que le budget européen, de 158 milliards, sera insuffisant pour répondre aux enjeux d'une Europe audacieuse, tels qu'ils ont été identifiés. Comme le soulignait il y a quelques jours Michel Barnier lors d'une audition au Sénat, le groupe centriste est convaincu que seule a cette masse critique et dispose d'une autorité légitime pour porter les valeurs de la France et ses intérêts dans le monde. Aussi voterons-nous ce budget. Mais, avant Mais, avant toute chose, il s'agit de bien négocier le du Brexit. À ce jour, les Vingt-Sept ont réussi à dépasser les flottements qui ont suivi l'annonce du Brexit et à échapper à une vague de populisme qui aurait pu balayer l'Europe, prouvant ainsi la solidité et même le regain de l'idéal européen. Ils sont aujourd'hui « unis

que le fait d'être membre à part entière. Pour conclure, je citerai une fois de plus notre négociateur : « Il y a une chose que j'ai comprise, c'est que ce que nous ne ferons pas ensemble, entre Européens, pour construire notre avenir, personne ne le fera à notre place. » Très bien ! La parole est à Mme Colette Mélot.

à examiner l'article 27 relatif à la participation de la France au budget de l'Union européenne. C'est un sujet de première importance, sachant que la France est le deuxième contributeur net européen après l'Allemagne, avec 19,1 milliards d'euros versés en 2017. Notre participation au budget européen représente ainsi 13 % de l'ensemble des contributions nationales. En retour, la France a touché 14,5 milliards d'euros de dépenses, soit 11 % des dotations accordées à des États membres. Notre pays est ainsi le premier bénéficiaire européen des dépenses de la politique agricole commune, avec une dotation européenne de 9 milliards d'euros. Il est également intéressant de noter que l'Union européenne abonde également les fonds français de politique de recherche et de développement, à hauteur de 2,221 milliards d'euros. En réalité, vous le savez, l'Union européenne redistribue la quasi-intégralité de ses moyens auprès des États membres. Seules 6 % des dépenses européennes sont effectivement consacrées au fonctionnement des institutions, essentiellement aux frais administratifs des trois institutions européennes. L'actualité brûlante des dernières années nous incite cependant à revoir rapidement notre stratégie d'affectation des crédits européens. Depuis plus de trente ans, des dirigeants de tous les pays européens appellent à renforcer le budget européen pour accroître nos capacités d'action. D'ailleurs, un groupe de travail planche depuis plus de trois ans sur la recherche de nouvelles ressources propres pour l'Union européenne. Dépenser davantage ensemble, c'est en effet conduire des économies, en limitant nos dépenses individuelles et en mutualisant nos actions. Il est plus que temps de donner à l'Union européenne les moyens d'agir. Le rapport Monti de janvier 2017 a ainsi tiré la sonnette d'alarme sur l'urgence de réformer le budget européen, tant sur les recettes que sur les dépenses. Ce besoin de repenser le budget européen n'est d'ailleurs pas une demande franco-française. Pour répondre à la crise économique et financière, puis à la crise migratoire, l'Union européenne a multiplié ces dernières années les fonds hors budget européen, comme le Mécanisme européen de stabilité créé en 2012. Deux défis méritent notre attention dans la réflexion sur la participation française au budget européen : la nouvelle politique européenne de défense et l'épreuve du Brexit. Sur la politique européenne de défense, 20 États membres ont signé, mercredi 8 novembre, un pacte de défense visant à créer un noyau dur de pays capables de financer et de faire vivre une vraie coopération militaire au niveau européen, avec la production de nouveaux matériels militaires, la mise en place d'une force commune d'intervention et l'établissement d'un budget européen de défense. Ces engagements, que nous soutenons fortement, s'inscrivent dans la continuité de la Coopération structurée permanente, la PESCO, signée en juillet dernier. des conséquences du Brexit sur le budget européen, il convient de rappeler que l'Union européenne perdra l'un de ses principaux contributeurs. Le départ du Royaume-Uni déclenchera ainsi une perte de recettes à court terme, avec l'arrêt du versement de sa contribution, soit une diminution de 6 % à 7 % du budget européen actuel. De nombreuses options sont encore sur la table, mais le doute subsiste sur l'avenir de l'équilibre financier de l'Union européenne. Il s'agira donc de s'assurer que le Royaume-Uni s'engage à respecter, coûte que coûte, ses engagements financiers conclus dans le cadre du cadre financier pluriannuel 2014-2020. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, face aux nouveaux défis de ce siècle, une action collective au plan européen est la seule solution viable. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires vous invite donc à envisager une participation plus ambitieuse de la France au projet européen, afin de doter l'Union européenne des moyens nécessaires à son développement. Nous souhaitons que le Gouvernement poursuive son engagement en ce sens.

Cette Europe réelle, charnelle, c'est une union des nations, une Europe qui, tout en reconnaissant ses dénominateurs communs, respecte chacun des peuples qui la composent et sont attachés à leur liberté et leur identité propre. On a beaucoup dévoyé la position du Front national sur l'Europe. Aussi, je le dis ici de façon claire et définitive, oui, nous sommes Européens ! De fait, que vous soyez, comme vos parents, né à Brest ou à Vladivostok, vous êtes Européen vous ne le serez jamais si vous résidez à Istanbul ! C'est précisément parce que nous sommes pour une Europe des nations libres et des peuples souverains que nous combattons cette Union « européiste », véritable machine à broyer les libertés, les souverainetés, les identités nationales. Un monstre froid, bureaucratique, technocratique, dogmatique qui ignore la volonté des peuples pour imposer une Europe de la finance, une Europe qui ne serait plus qu'un terrain de jeu pour le nomadisme économique et migratoire. Quand, de Paris à Londres, en passant par Vienne, Varsovie, Budapest, Amsterdam et même Berlin, les peuples se lèvent pour dire non à votre Europe antidémocratique, quelle est votre réponse ? Une incarcération européenne plus dure encore, décidée par les geôliers de la Commission de Bruxelles et la Cour européenne des droits de l'homme- des droits de l'homme, mais jamais du citoyen ! Or la réalité européiste est accablante : la politique européenne de défense est une chimère ; la politique agricole commune a ruiné notre agriculture la directive sur les travailleurs détachés est un véritable fléau et l'opération d'agitprop d'Emmanuel Macron, largement relayée par des médias complaisants, n'y changera rien, puisque le nombre de ces travailleurs dépasse désormais

Afin de faire disparaître les États-nations, l'Union européenne encourage l'émergence de grandes régions capables de passer outre le niveau étatique. Cette stratégie de désintégration nationale n'est pas sans responsabilité dans la crise que subit aujourd'hui l'Espagne. Depuis plusieurs années, notre contribution au budget de l'Union européenne est en constante augmentation.

L'Europe, c'est le berceau de la civilisation occidentale, helléno-chrétienne. C'est un héritage, un équilibre, un assemblage de nations qui aspirent à coopérer, tout en préservant leur liberté. Nous ne saurions dès lors cautionner une telle soumission à la vieille construction européiste,

ce qui nous protège et ce qui nous donne un avenir ». Je partage cette vision, qui nous éloigne d'une Europe comptable. Mais l'examen de ce jour sur le prélèvement européen des recettes de l'État, fixé à 20,2 milliards d'euros pour 2018, nous invite immanquablement à une approche plus terre à terre. Comme on pourrait le dire plus familièrement au regard de notre contribution, en avons-nous pour notre argent ? Nous connaissons l'équation, notre rapporteur spécial l'a d'ailleurs brillamment détaillée la France est le deuxième contributeur net, en volume, au budget de l'Union européenne, derrière l'Allemagne, tout en étant le troisième bénéficiaire des politiques européennes. Notre pays profite en particulier des deux principaux instruments d'investissement de l'Union européenne : la politique agricole commune et le Fonds européen pour les investissements stratégiques. de la PAC, nos agriculteurs percevront 9 milliards d'euros en 2018, soit la moitié, environ, de notre contribution. Cela dit, je m'inquiète de la diminution des soutiens européens au cours des derniers exercices budgétaires. Cette baisse est le fruit de l'actuelle programmation financière pluriannuelle de l'Union européenne et jette un doute sur la volonté de maintenir la PAC comme une priorité. Madame la ministre, vous connaissez la situation difficile que traversent beaucoup d'agriculteurs. Nous devons pouvoir compter sur vous pour que l'agriculture européenne soit confortée dans le cadre financier pluriannuel post-2020. La politique agricole commune doit demeurer une priorité de la politique communautaire. S'agissant du Fonds européen pour les investissements stratégiques, le bilan tiré de la première phase arrêtée en 2016 a démontré que notre pays était le principal bénéficiaire du plan Juncker, avec 15 milliards d'euros. Nous devons nous en féliciter. Nous pouvons ajouter à cette logique de « juste retour » des externalités positives non quantifiables, telle l'appartenance à un marché unique. Il n'est alors plus besoin de démontrer que nous ne devons jamais douter de l'Europe. Toutefois, mes chers collègues, ces points positifs pour la France n'exonèrent pas d'une réflexion sur l'architecture et le niveau des ressources européennes, réflexion rendue plus pressante à l'approche de la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. À terme, nous le savons, le Brexit privera le budget européen de 10 milliards d'euros. Des travaux ont été menés, notamment par le groupe de haut niveau sur les ressources propres. Un consensus existe sur la nécessité d'avoir des recettes plus lisibles, plus transparentes et plus équitables. Je tiens d'ailleurs à souligner la nécessité de mettre fin aux rabais et aux corrections, qui faussent les règles de solidarité, une valeur pourtant au coeur du projet européen. Il me semble également nécessaire d'instituer un cadre financier plus souple, afin de répondre, aux côtés des politiques traditionnelles, à la montée en puissance de certains enjeux : sécurité, lutte contre le terrorisme, gestion des flux de réfugiés et de migrants ou enjeux de défense- des opérations extérieures Dans les situations d'urgence, l'Union européenne a pu actionner les mécanismes de flexibilité dont elle disposait pour doubler les crédits. Mais on a aussi vu se développer, en parallèle, des mécanismes hors budget. Une part plus importante de budget non affecté pourrait donc être envisagée dans le prochain cadre pluriannuel. Plus précisément, sur la défense- je souhaiterais terminer mon l'effort demandé sera croissant compte tenu du contexte international actuel. Le Fonds européen de la défense, annoncé par la Commission européenne en juin dernier, est une bonne initiative. C'est un pas de plus vers l'Europe de la défense, même s'il reste encore un long chemin à parcourir. En attendant, il faudra encore compter sur l'engagement et le sens des responsabilités de certains États membres, au premier rang desquels la France, qui assume bien souvent, aux côtés du Royaume-Uni, l'essentiel des déploiements militaires extérieurs. Aussi, dans le cadre des discussions sur la contribution de chacun au budget européen, je pense qu'il serait opportun de prendre en compte le coût des engagements nationaux fournis par les États membres pour assurer la sécurité de l'Europe, engagements pour lesquels leur contribution est Mes chers collègues, le RDSE a eu l'honneur de compter parmi ses membres l'illustre Maurice Faure, cher à notre président de groupe Jean-Claude Requier, pour qui l'Europe était une idée, un esprit, une communauté de valeurs, mais aussi une réponse à des situations géopolitiques successivement L'élu de la Meuse que je suis en est pleinement conscient. Sachons nous mobiliser pour assurer l'avenir de l'Europe ! Nous voterons donc, madame la ministre, Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le montant du financement de la France à l'Union européenne pour l'année 2018. Cet exercice, je le rappelle, est très contraint puisqu'il s'inscrit dans le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, qui court de 2014 à 2020, alors que s'engagent d'ores et déjà les discussions pour le prochain cadre financier pluriannuel post-2020.

Pour notre pays, le montant du prélèvement sur recettes européen est estimé à 20,2 milliards d'euros pour 2018, contre 17,9 milliards d'euros en 2017. C'est un effort important, puisqu'il s'agit du quatrième poste du budget de l'État. Le budget européen doit aujourd'hui répondre à trois exigences : relever les défis ponctuels, préserver les politiques qui font l'identité de l'Union européenne et lancer de nouveaux projets communs. Parmi les défis à relever, la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la sécurité sont devenus une priorité depuis les attentats ayant frappé nombre de pays de l'Union européenne. Je ne reviendrai pas en détail sur l'ensemble des mesures prises qui, si elles sont encore insuffisantes, vont tout de même dans le bon sens.

Cette prise de conscience récente d'une politique commune en matière de sécurité, comme en matière de migration, a bien évidemment un coût, qui n'était pas forcément anticipé dans le cadre financier pluriannuel actuel. La Commission européenne a toutefois mobilisé les crédits nécessaires, faisant preuve- c'est assez nouveau pour être signalé -de pragmatisme et de souplesse, même s'il convient d'être vigilant sur la réaffectation de crédits dont pourraient souffrir d'autres politiques de l'Union D'ailleurs, au-delà de la question des mécanismes de financement du budget européen, l'introduction de plus de souplesse et la simplification de l'exécution budgétaire sont indispensables. On ne peut plus continuer avec un cadre budgétaire pluriannuel aussi rigide, car, au contexte budgétaire délicat que connaissent à la fois l'Europe et les pays membres, s'ajoute un système d'exécution particulièrement lourd et archaïque. Ainsi, à l'occasion de la révision à mi-parcours du cadre financier actuel, les instruments de flexibilité ont dû être débloqués au maximum. Il a fallu batailler pour préserver le financement de politiques pourtant considérées, dans les discours, comme prioritaires. Cette mauvaise prévisibilité a eu entre autres conséquences une multiplication des budgets rectificatifs- déjà six

L'Europe doit bien évidemment être une « assurance stabilité », et il est souvent positif de programmer telle ou telle politique sur le long terme. Mais l'Europe doit aussi être capable de réagir vite et de façon massive. Elle est aujourd'hui soumise à des aléas d'ordre financier, économique, climatique, géopolitique et social qu'il faut être en mesure de traiter. La hausse de la dotation de l'initiative pour l'emploi des jeunes, pour la porter à un total de 600 millions d'euros, ou encore la montée en puissance du plan Juncker sont de ce point de vue tout à fait satisfaisantes. Rapprocher l'Europe et le citoyen, c'est avant tout construire une Europe dynamique, qui protège les citoyens européens. Bref, aussi bien pour le financement que pour l'exécution budgétaire, il est temps de changer le logiciel. La négociation du futur cadre budgétaire post-2020 sera ainsi abordée dans un contexte budgétaire délicat. Il n'y aura pas d'issue sans argent frais ! Plusieurs scénarios sont proposés, en particulier par le groupe présidé par Mario Monti, qui a réfléchi pour trouver des moyens de financement plus transparents, simples, équitables et démocratiquement responsables. Il est peut-être temps de passer à l'action pour doter l'Union européenne de nouvelles ressources propres. Malheureusement, nous l'affirmons chaque année avec une force croissante, mais sans grand succès. La question budgétaire est au coeur de la refondation de l'Union européenne : il faut mettre en adéquation les financements avec les ambitions. Ce budget doit en être le signal.

de la politique de cohésion, deux éléments suscitent l'inquiétude : d'une part, la sous-consommation des crédits actuels déjà évoquée et, d'autre part, les pistes de réforme pour la période postérieure à 2020. Au milieu de l'année 2017, moins de 10 % des crédits d'engagement de la politique de cohésion avaient donné lieu à des paiements,

L'autre sujet d'inquiétude dans ce domaine concerne le septième rapport sur la cohésion adopté par la Commission européenne le 9 octobre dernier. Cette dernière n'a pas hésité à lancer des pistes de réformes, qui conduiraient à de grands bouleversements fin de la couverture intégrale du territoire européen, renforcement des conditionnalités d'attribution des fonds structurels et d'investissement, mise en place d'un fonds unique d'investissement, augmentation des taux de cofinancement nationaux, comme pour la PAC d'ailleurs, régionalisation des recommandations pays par pays dans le cadre du semestre européen, création d'un nouveau fonds pour soutenir les réformes structurelles. Elle prévoit également la possibilité d'une introduction de nouveaux critères dans l'attribution des enveloppes budgétaires. Ce serait alors la victoire de ceux qui essaient, depuis des années, d'introduire ce système de conditionnalités, contre l'avis de la France. Plusieurs organisations européennes représentant les collectivités locales et régionales se sont inquiétées, à juste titre, de ces pistes de réflexion. Nous devons appeler à la mobilisation de toutes et tous pour sauver la politique de cohésion, et même pour encourager son amplification. il ne faudrait pas que, à une politique de subventions, soit substituée une politique de prêts garantis. C'est un changement de doctrine qui apparaît en filigrane dans certaines politiques de l'Union Prenons l'exemple d'Erasmus et Erasmus+, qui permettent l'octroi de bourses d'études : certains ici ou là souhaiteraient que le fonctionnement de ces dispositifs soit calqué sur le plan Juncker et que, à la place de bourses, les étudiants aient accès à des prêts avantageux. Il faut veiller à ce que l'Union européenne ne multiplie pas les dispositifs de prêts, qui vont, pour le coup, plus en direction du secteur privé et moins en direction du secteur public. Pour notre part, nous serons vigilants et intransigeants sur ce point particulier. Nous souhaitons qu'elle puisse se réformer pour être plus réactive et en phase avec les défis contemporains. Nous souhaitons qu'elle puisse répondre aux attentes des citoyens européens. Nous souhaitons tout simplement qu'elle réussisse.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'examen de la contribution française au budget de l'Union européenne est un moment fort du débat parlementaire consacré à l'Europe. Celui que nous menons aujourd'hui ne fait pas exception à la règle, et, à la lumière des éléments apportés par le rapporteur spécial de la commission des finances, le groupe Les Républicains votera en faveur du prélèvement sur recettes tel qu'il est proposé. Mais nos discussions revêtent cette année une dimension supplémentaire, puisqu'elles entrent en résonance avec le débat sur la refondation de l'Europe. En effet, la mue que l'Union européenne va devoir opérer ne saurait se satisfaire d'un budgétaire. Très clairement, le prochain cadre financier pluriannuel, dont les premiers contours seront présentés en mai 2018, devra faire face à d'importants défis. Le premier d'entre eux est bien évidemment le Brexit. Au-delà des négociations sur la facture dont le Royaume-Uni devra bien sûr s'acquitter à son départ, le Brexit entraînera un manque à gagner d'environ 10 milliards d'euros par an pour le budget européen. Par ailleurs, un certain consensus semble se dessiner sur la nécessité d'une action commune dans le domaine des « nouvelles priorités » que sont la défense, la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ou encore la gestion des frontières extérieures et des migrations. S'il faut à mon sens s'en féliciter, il n'en reste pas moins que les ambitions affichées devront se matérialiser par des niveaux de financement crédibles, comme cela est proposé, par exemple, dans le domaine de la défense l'initiative d'un fonds européen spécifique. Selon la Commission européenne, le besoin de financement découlant de ces priorités se chiffrerait à 10 milliards, voire à 15 milliards d'euros par an. Sans même évoquer la question des différents projets de budgets spécifiques à la zone euro ou celle des crédits accordés à d'autres objectifs politiques majeurs, ce serait donc, au bas mot, 20 milliards à 25 milliards d'euros annuels qu'il faudrait trouver. Si l'on s'en tient, comme cela me semble souhaitable, à l'impossibilité pour l'Union européenne d'émettre de la dette, la solution de cette équation ne peut donc passer que par deux leviers : d'une part, une réduction des dépenses et, d'autre part, une augmentation des recettes. S'agissant des dépenses, permettez-moi tout d'abord d'insister sur la nécessité de leur passage en revue systématique à l'aune des principes de subsidiarité et d'efficacité. En effet, si l'Europe n'a pas vocation à régenter les détails de notre vie quotidienne, elle n'a pas non plus vocation à financer ce qui relève à l'évidence de l'action nationale, voire locale. La clarification que nous devrons mener sur la répartition des compétences entre l'Europe et les États membres devra ainsi trouver son corollaire au niveau budgétaire, en recentrant les financements communautaires sur l'ensemble des défis communs. Chaque euro dépensé devra faire la preuve de sa valeur ajoutée, c'est-à-dire être investi dans des domaines et des projets pour lesquels l'action européenne n'est pas seulement appropriée, mais indispensable et, surtout, efficace. À cette fin, une « culture d'évaluation de la dépense » doit se faire jour au niveau européen, en miroir de l'évaluation législative désormais à l'oeuvre. Mais nous devons également avoir à l'esprit que la réflexion sur les dépenses accentuera nécessairement la pression sur la politique de cohésion et la politique agricole commune, ces dernières représentant les deux tiers du budget. Si l'on souhaite préserver autant que possible leur financement- tout particulièrement celui de la PAC, à laquelle mon groupe est profondément attaché -, il faudra les faire évoluer.

Pour notre pays, contributeur net dont le prélèvement sur recettes représente tout de même le quatrième poste de dépenses de l'État, cela constituerait un effort supplémentaire non négligeable. Dès lors, et même si je suis convaincu que le budget de l'Union européenne est bien plus qu'un simple jeu à somme nulle opposant des contributeurs à des bénéficiaires, il faudra à mon sens engager une réflexion sur la manière de prendre en compte la participation des contributeurs nets dans le calcul de leurs déficits publics. En effet, il serait pour le moins difficile de comprendre qu'une contribution française en hausse significative puisse éventuellement se traduire par des difficultés à respecter les critères du pacte de stabilité et de croissance. Par ailleurs, comment accepter une pression accrue sur nos finances publiques si celle-ci ne s'accompagne pas, enfin, de la suppression définitive de tous les rabais et autres corrections dont bénéficient plusieurs États membres ? Cette réforme ne peut plus être repoussée, car il en va non seulement de la transparence sur les ressources de l'Union européenne, mais également du principe d'équité entre les États membres. En tout état En tout état de cause, ces éléments montrent bien à quel point il serait malaisé de mobiliser encore davantage les contributions directes issues des budgets nationaux. Bien que ce sujet soit indéniablement sensible, le temps paraît ainsi venu de donner plus de place à des ressources véritablement propres. De nombreuses propositions ont d'ores et déjà été avancées en la matière. Il me semble néanmoins que plusieurs principes, dont certains ont d'ailleurs été rappelés par le groupe de haut niveau présidé par Mario Monti, doivent guider notre réflexion. Tout d'abord, je crois que l'Union européenne devrait se pencher prioritairement sur la ressource TVA existante. Celle-ci pourrait contribuer beaucoup plus au financement de l'Union européenne, en particulier si la lutte contre la fraude- estimée à 150 milliards d'euros par an - et, plus largement, la lutte contre l'évasion fiscale étaient rendues plus efficaces. Ensuite, rappelons que les ressources propres ne peuvent être assimilées à des taxes européennes, car le pouvoir fiscal est, et doit bien évidemment demeurer, du ressort national. Par ailleurs, le but ne doit pas être en soi d'augmenter automatiquement le budget européen, dont le volume adéquat doit faire l'objet d'un débat spécifique. L'objectif premier doit bien être de modifier la composition des recettes qui l'alimentent et, donc, de contribuer à stabiliser, voire à réduire les contributions directes des États membres. La réforme du financement de l'Union européenne ne devra pas non plus conduire à alourdir l'imposition des citoyens. De ce fait, chaque euro prélevé au bénéfice de l'Union européenne devra diminuer d'autant la charge fiscale au niveau national. Il sera en outre indispensable de veiller à ne pas plomber la compétitivité européenne en asphyxiant la production, et donc privilégier les options qui seront au contraire de nature à la conforter, comme, par exemple, l'instauration d'une taxe carbone aux frontières ou, plus largement, de taxes antidumping robustes. Enfin, de telles évolutions rendront encore plus indispensable, selon moi, une implication accrue des parlements nationaux dans le processus de décision budgétaire, notamment lorsqu'il s'agira de définir des ressources propres, d'adopter le cadre financier pluriannuel ou de contrôler l'exécution du budget de l'Union Madame la ministre, mes chers collègues, vous l'aurez constaté, si le vote du groupe Les Républicains en faveur du prélèvement sur recettes marque sa volonté de donner à l'Europe les moyens de réaliser les objectifs que nous lui assignons, il n'en est pas moins l'expression

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires européennes, monsieur le vice-président de la commission des finances, monsieur le rapporteur spécial, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite tout d'abord vous remercier pour ce débat c'est un moment démocratique important pour évoquer la contribution de la France au budget commun et ce qu'elle en retire, mais aussi pour mettre l'accent sur la valeur ajoutée des politiques que nous menons ensemble, au niveau européen.

qui s'élèvera donc à 160,1 milliards d'euros au titre des crédits d'engagement et à 144,7 milliards d'euros au titre des crédits de paiement. Cela respecte les objectifs que nous nous étions fixés en termes de marge sous plafond. Les services du ministère de l'action et des comptes publics en étudient actuellement l'impact sur l'estimation de notre prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne pour 2018. En ligne avec nos priorités européennes, ce budget, qui doit encore être formellement adopté par les deux institutions d'ici à la fin du mois, permettra de dégager les financements nécessaires pour la croissance, l'investissement, l'emploi- oui, monsieur Ouzoulias, ce sont bien là nos préoccupations prioritaires, et aujourd'hui, l'ensemble de la zone euro a renoué avec la croissance et les mesures en faveur de la jeunesse, qui en sont les principales priorités, avec, notamment, une montée en charge sur les programmes comme Erasmus+, ainsi que vous l'avez, à juste titre, relevé, monsieur et un renforcement des moyens du Fonds européen pour les investissements stratégiques, établi dans le cadre du plan Juncker, dont vous avez parlé, monsieur Menonville. Nous y avons veillé, les montants dédiés à la croissance et l'emploi ont globalement été accrus par rapport à la proposition initiale de la Commission. Ce budget permettra aussi le renforcement des moyens destinés à l'aide humanitaire et la poursuite de la montée en puissance de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

et pour mettre en réserve d'autres crédits destinés à ce pays, à hauteur de 70 millions d'euros en crédits d'engagement et 35 millions d'euros en crédits de paiement, qui seront mobilisables en fonction de la situation de l'État de droit, de la démocratie, des droits de l'homme et de la liberté de la presse. Je viens de revenir brièvement sur les grands paramètres des dépenses du budget 2018. Pour appréhender le montant du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne, il est légitime de chercher à nous situer par rapport aux autres États membres. Plusieurs d'entre vous l'ont relevé, la France est le deuxième contributeur net en volume, après l'Allemagne. Notre solde net est de fait négatif, bien entendu, et nous l'assumons, monsieur Car il est avant tout l'expression du fait que nous sommes dans le groupe des « pays moteurs » de l'Union, et que nous exprimons notre solidarité envers nos partenaires en rattrapage économique et dont on oublie encore trop souvent d'où ils viennent. Nous concentrer uniquement sur ce solde net présenterait néanmoins le risque de réduire notre débat à un chiffre qui ne permet en aucun cas de prendre la juste mesure de l'ensemble des bénéfices que nous retirons de notre appartenance à l'Union européenne en premier lieu, faire partie d'un grand marché unique de 500 millions d'Européens, dont nos entreprises tirent chaque jour profit. Nos amis britanniques en font d'ailleurs l'amère expérience en mesurant, au fil des annonces des opérateurs économiques qui envisagent de quitter le Royaume-Uni, les conséquences de leur sortie prochaine. S'agissant du Brexit, je souhaite souligner que son impact sur le budget européen sera nul pour l'année à venir. Quant aux budgets suivants, tout dépendra de l'issue des négociations en cours entre l'Union européenne et le Royaume-Uni en ce qui concerne le règlement financier dont devra s'acquitter Londres au titre des engagements souscrits en tant que membre de l'Union européenne. Dans l'hypothèse d'un Brexit, et si le Royaume-Uni cessait brusquement toute contribution, l'impact budgétaire serait majeur dès 2019. On ne peut écarter ce scénario, même si nous travaillons activement pour que la raison prévale. Au-delà, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne entraînera le départ d'un important contributeur au budget européen, ce qui pèsera sur le prochain cadre financier pluriannuel pour l'après-2020, comme l'ont rappelé le président Bizet et Mme Mélot. Parmi l'ensemble des défis auxquels l'Europe est confrontée, de nouvelles priorités sont par ailleurs apparues ou montent en puissance, comme la défense, la sécurité ou bien La révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2014-2020 a permis quelques premières avancées en ce sens. Ces nouvelles priorités devront donc être prises en compte dans les prochaines perspectives financières de l'Union, tandis que d'autres politiques plus traditionnelles, comme la politique agricole commune et la politique de cohésion, que vous êtes nombreux à avoir mentionnées, resteront pleinement d'actualité. Plus que réviser à la marge ces politiques sous contrainte budgétaire, nous devons, de façon équilibrée, procéder à des transformations de fond dans le respect de nos intérêts. Le Président de la République l'a dit, par exemple, au sujet de la PAC, monsieur Cuypers, monsieur Menonville, madame Loisier. Celle-ci doit être rénovée pour devenir « l'instrument de la transition agricole, de notre souveraineté, face aux grands défis de la mondialisation ». Nous y travaillons avec le ministère de l'agriculture et l'ensemble des ministères concernés. Concernant la politique de cohésion, monsieur Sutour, n'ayons pas peur des mots, ni de réfléchir

Cohésion veut dire convergence. Parmi les nouvelles priorités de l'Union européenne, vous l'avez évoqué, madame Mélot, monsieur Menonville, celle de l'Europe de la défense est en train de devenir une réalité politique. Nous progressons sur le Fonds européen de la défense. Vingt-trois États membres ont notifié officiellement lors du dernier conseil Affaires étrangères du 13 novembre leur intention de participer à la coopération structurée permanente, qui devrait être lancée en décembre. Bien sûr, du point de vue budgétaire, nous n'en sommes qu'au tout début. C'est dans le prochain cadre financier que l'effort sera véritablement à faire. Je voudrais malgré tout mentionner deux aspects concrets qui relèvent des budgets pour 2018 et 2019. Tout d'abord, l'action préparatoire sur la recherche en matière en matière de défense, finance, à hauteur de 90 millions d'euros entre 2017 et 2019, dont 40 millions en 2018, des projets de recherche qui ne pourraient pas être financés dans le cadre du programme de recherche européen Horizon 2020. Cette action préfigure le volet « recherche » du Fonds européen de la défense, dont nous souhaitons le lancement au début de 2018. Ce fonds comportera également un volet destiné au développement de capacités, qui s'inscrira dans le prolongement du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, proposé par la Commission et qui devrait pouvoir financer des premiers projets dès 2019. Ensuite, plus largement, permettez-moi de souligner que, si le départ britannique est une contrainte forte, il est aussi une opportunité de repenser le budget européen au regard de nos priorités politiques. Et cela est vrai des dépenses comme des recettes. S'agissant de ce second volet, la sortie du Royaume-Uni représente une occasion historique de remettre à plat le système de financement du budget européen. La France a d'ailleurs accueilli favorablement le rapport final du groupe de haut niveau sur les ressources propres, présidé par Mario Monti, que vous avez mentionné, monsieur le rapporteur spécial, monsieur Sutour, et attend avec intérêt l'examen à venir par la Commission des pistes de nouvelles ressources propres envisagées. En tout état de cause, le départ du Royaume-Uni entraîne mécaniquement la disparition du rabais britannique, et la France soutient en conséquence la disparition de l'ensemble des chèques et des rabais dont quelques contributeurs bénéficient, contrairement à nous- vous avez raison, monsieur À terme, nous avons également pour objectif la création d'un budget pour la zone euro, qui financera des investissements et sera doté d'une fonction de stabilisation. Parmi les pistes de ressources envisageables pour financer celui-ci, le Président de la République a évoqué dans son discours de la Sorbonne des taxes européennes dans le domaine du numérique ou de l'environnement, ou bien encore l'affectation de la fraction d'un impôt à ce budget, par exemple l'impôt sur les sociétés, une fois son harmonisation réalisée. Je souligne d'ailleurs que nous portons l'ambition commune avec l'Allemagne de parvenir dans les quatre prochaines années à l'harmonisation des bases de l'impôt sur les sociétés. En outre, la France a proposé une feuille de route européenne sur la fiscalité du numérique. Après le Conseil européen d'octobre, une proposition législative de la Commission est attendue au début de 2018. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, après le discours de la Sorbonne du Président de la République et les débats que nous avons eus dans cet hémicycle sur l'avenir de l'Union européenne, la question qui m'amène aujourd'hui est bien plus immédiate au nom du Gouvernement, je vous demande en effet d'autoriser le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne pour l'année 2018. Pour conclure, je voudrais souligner combien cette contribution est fondamentale seulement pour l'équilibre du budget européen pour 2018, mais aussi parce qu'elle exprime notre adhésion à la construction européenne, notre volonté d'agir ensemble et de pouvoir tirer profit ensemble des bénéfices qu'apporte la participation au plus grand marché unique et à la plus puissante zone commerciale intégrée au monde, comme vous l'avez rappelé, monsieur Gattolin. Bien évidemment, la construction européenne crée aussi des frustrations et des insatisfactions. Je gage que nous ne sommes pas forcément tous d'accord sur la meilleure manière de refonder l'Europe. Ces divergences sont légitimes. C'est la raison pour laquelle le Président de la République souhaite, parallèlement au processus de refondation de l'Europe, l'organisation de conventions démocratiques, qui permettront d'écouter les citoyens européens sur ce que l'Union fait bien, trop peu, trop, ou trop difficilement. Je sais pouvoir compter sur le Sénat pour participer à cette réflexion. Il reste cependant, et c'est là l'essentiel, que notre contribution nationale au budget européen marque notre engagement européen. Nous avons bien la conviction que c'est à l'échelle de l'Europe que nous pourrons au mieux garantir notre souveraineté. Je vous remercie, et je reste à la disposition du Sénat.

qu'on imagine et que je ne développerai pas ici. Selon nous, il faut interroger le projet européen libéral de concurrence libre et non faussée. C'est l'occasion de le faire, de prolonger un peu le débat que nous venons d'avoir. C'est une Europe qui inquiète, on le sait, une Europe qui divise, une Europe qui oppose tout le monde à tout le monde, malheureusement, c'est l'Europe du social et fiscal que l'on a déjà évoquée. Ce sont là des questions de fond. La question se pose singulièrement : quelle destination pour cette contribution financière au projet européen ? Alors oui, parlons de l'Europe. Nous, nous voulons changer cette Europe- contrairement à ce que entend souvent, les communistes seraient, de toute façon et par principe, contre l'Europe ! -, nous sommes pour une Europe humaniste, une Europe de la coopération mutuellement avantageuse entre les nations et les peuples, une Europe de la paix

ces engagements. C'est pourquoi il est nécessaire de doter l'Europe des moyens lui permettant d'agir. En même temps, on sait bien qu'un certain nombre de problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne pourront se régler que par une meilleure coopération entre les différents pays européens.